Monsieur le ministre, mes chers collègues,

que nous avons appris, le 3 mars dernier, la disparition de notre collègue Alain Bertrand, sénateur de la Lozère, qui nous a quittés à l'âge de 69 ans, après avoir mené pendant de longs mois un combat courageux et digne contre la maladie. Nous étions présents à ses obsèques,

Ce fut une émouvante cérémonie d'adieu, à laquelle assistaient nombre d'habitants de la Lozère et de personnalités politiques et d'élus de son département. Didier Guillaume, présent aujourd'hui et que je salue, lui a rendu un hommage empreint à la fois d'affection profonde et de grand respect.

Loire. Il en fut l'ardent avocat dans notre hémicycle tout au long de ses dix années de mandat. Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue fortement impliqué dans le travail parlementaire, particulièrement sur les questions concernant l'aménagement du territoire et l'agriculture, mais aussi aussi d'un élu de terrain très attaché à son territoire et d'une personnalité chaleureuse, affable et pleine d'humour. d'humour. Né le 23 février 1951 à Saint-Juéry dans le Tarn, Alain Bertrand avait choisi la profession d'inspecteur des domaines après des études à l'École nationale des finances publiques de Clermont-Ferrand. Il se fixa dans le département de la Lozère, qui devint sa terre d'adoption. C'est là qu'il s'engagea en politique en adhérant au parti socialiste, dont il devint premier secrétaire de la fédération départementale, et qu'il exerça de nombreux mandats locaux. Il siégea au conseil régional du Languedoc-Roussillon de 1998 à 2011 et en devint à la fois vice-président et président de la commission « Montagne-élevage, chasse et pêche » de 2004 à 2011. À partir de 2001, il fut aussi conseiller municipal de Mende, puis maire de cette ville de 2008 à 2016. Au cours de cette période, il fut également président de la communauté de communes Coeur de Lozère. Alain Bertrand a largement marqué de son empreinte la ville de Mende. Ainsi est-il à l'origine de bien des réalisations locales : il s'est notamment beaucoup investi pour doter l'hôpital de Mende Lozère des équipements les plus modernes. 2011, Alain Bertrand fit son entrée au Sénat, devenant le premier sénateur de gauche du département de la Lozère depuis la Seconde Guerre mondiale. Réélu lors des élections sénatoriales de 2017, il se consacra alors prioritairement à son mandat sénatorial. Il avait en effet choisi de conserver son mandat de sénateur « pour pour défendre fidèlement les intérêts de toute la Lozère ». Au Sénat, c'était un membre particulièrement actif de la commission des affaires économiques, dont il était vice-président depuis 2014, après avoir été vice-président de la commission des affaires européennes. Il intervenait très régulièrement, en commission comme en séance, dans les débats concernant notamment l'aménagement du territoire et l'agriculture. Alain Bertrand s'était en particulier illustré par son combat pour cantonner la présence du loup dans les seuls territoires inhabitables, considérant que le retour de ce grand prédateur semait le trouble et l'insécurité des biens et des personnes dans les campagnes, attaché qu'il était aussi au pastoralisme et à l'élevage. La proposition de loi qu'il déposa, tendant à créer des « zones d'exclusion totale » au sein desquelles la présence du loup serait déclarée indésirable, répondait à ce dessein. Ce texte fut adopté ici même en 2013, et certaines de ses dispositions furent prises en compte par le Gouvernement dans le cadre du plan Loup 2013-2017. En 2014, Alain Bertrand fut chargé par le gouvernement d'alors d'une mission temporaire sur les territoires hyper-ruraux qui a donné lieu à un rapport remarqué, dans lequel notre ancien collègue mettait l'accent sur la situation « critique, voire au seuil de l'effondrement » de ces territoires ... Selon lui- je cite les conclusions de son rapport -, « il ne peut y avoir de sous-territoire, de même qu'il ne peut y avoir de sous-citoyen et de minorité sacrifiée et interdite d'avenir au profit ... non pas tant du bien-être de la majorité, mais plutôt du seul respect d'une vision dominante, nourrie par les habitudes, les indicateurs et la mécanique des processus de décision. « La solidarité républicaine et la cohésion nationale doivent donc l'emporter,

formulait-il des propositions originales en ce sens, comme la création d'un « guichet unique hyper-ruralité » pour favoriser les initiatives, un droit à pérennisation pour les expérimentations efficientes

Ces propositions ont permis l'éveil d'une prise de conscience au sein de l'exécutif. Des progrès ont été réalisés. Il reste encore beaucoup à faire. La voix d'Alain Bertrand nous manque. La leçon de ce jour est aussi de rester fidèle au message qu'il a su porter ici avec tant de passion. Au-delà de sa carrière politique brillante, de sa grande maîtrise de ses dossiers, de sa connaissance profonde du terrain, Alain Bertrand laissera le souvenir d'un homme convivial et bon vivant, amateur de rugby et de football. Il avait une prédilection particulière pour la pêche- je puis le comprendre ... Il fut ainsi longtemps- je n'ai jamais accédé à cette dignité ! -président de la Fédération de pêche de son département. Cette activité, comme la chasse, le plongeait dans la nature riche et diverse et dans la beauté des paysages de la Lozère, dont il était si familier. Je tiens à rendre hommage à ses qualités humaines et à saluer son empathie, sa générosité, son attention aux autres. Oui, il aimait la Lozère, et il aimait encore plus ses habitants, dont il aura défendu inlassablement les intérêts. Au-delà, il s'était engagé sans compter pour que des réponses adaptées soient apportées aux difficultés spécifiques des habitants de ces territoires si chers à son coeur. À ses anciens collègues des commissions des affaires économiques et des affaires européennes, à ses amis du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, j'exprime de nouveau notre sympathie. À toute sa famille, à ses proches, à ses collègues qui lui ont succédé à Mende, à tous ceux à qui il était cher et qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire, en ce moment de partage et de recueillement, la part que le Sénat continue de prendre à leur deuil. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille ... Le courage, c'est d'aller à l'idéal », écrivait Jean Jaurès, qu'il admirait tant. Alain Bertrand a profondément aimé la vie. Sans doute a-t-il affronté la mort d'un regard tranquille ; nous sommes certains qu'il est aujourd'hui allé à l'idéal que décrivait Jean Jaurès. Monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice de Lozère, chère Guylène Pantel, monsieur le maire de Mende, cher Laurent, madame la présidente du département, mesdames, messieurs les membres de la famille, vous l'avez rappelé, monsieur le président, nous étions présents, avec la présidente Primas, avec le président Requier et avec de très nombreux autres élus, le 6 mars dernier, pour rendre un dernier hommage à Alain Bertrand.

hommage à un élu de la Nation, à un républicain atypique et attachant, à un homme, tout simplement. Le Gouvernement s'associe à l'hommage que vous venez de lui rendre, monsieur le président, un hommage- cela n'étonnera personne -plein de sincérité, d'amitié et de vérité.

Je m'imagine parfois comment Alain Bertrand, cet homme de dialogue et d'ouverture, aurait pu traverser cette période de deux mois et demi, lui qui ne vivait jamais aussi bien que dehors, au bord des cours d'eau, dans la forêt ou dans la montagne Je me plais à penser que le bon sens qui le caractérisait nous aurait montré la voie, sans perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, pour ce genre d'homme, c'est de savoir d'où l'on vient, pour comprendre où l'on va.

Pour lui, les choses sont claires : aucun poste de haut fonctionnaire ne saurait être une source de bonheur équivalente à une vie en Lozère. Il s'y établira et ne la quittera plus. Alain Bertrand fait de ce département son terrain de jeu et son terrain d'engagement politique. Il aimait raconter que, à la sortie d'une réunion publique, à Mende, il s'était précipité dans une cabine téléphonique pour appeler son père et lui dire : « J'ai rencontré un véritable leader politique, un visionnaire érudit d'une intelligence rare. Il voit loin et juste, et il est Tarnais ». Cet homme, c'était Georges Frêche,

Je ne reviendrai pas sur son parcours politique, long et difficile dans cette terre lozérienne- vous l'avez très bien fait, monsieur le président -, mais je retiendrai deux événements. Tout d'abord, le courage et la ténacité dont il fit preuve pour devenir maire de Mende en 2008. Une élection difficile, une victoire historique, une confiance renouvelée par ses amis administrés et un acquis solide revendiqué par l'actuelle équipe municipale, qui poursuit son oeuvre- je veux saluer Laurent Suau, son successeur

Pensez donc : ces deux hommes du terroir lancés face à face. Une bataille frontale d'hommes rusés, d'hommes forts, d'hommes aux forts accents. Âmes sensibles s'abstenir ! Je me souviens- je ne

Je veux également saluer la mémoire d'un homme, son engagement social, socle de ses convictions politiques les plus fortes, et surtout son engagement en faveur de la ruralité, de l'hyper-ruralité, source inépuisable d'idées pour apporter un nouvel élan à nos campagnes.

que les questions fondamentales de l'unité républicaine et de la vie commune se posent aussi dans la ruralité et dans l'hyper-ruralité ? Il ne faut jamais oublier les habitants de toute la France, de tous les territoires, les grands comme les plus petits.

toujours chronophages, il y avait l'homme. Il chérissait sa famille, sa fille Sylvie. Il aurait tant aimé connaître Pablo, son petit-fils, né à peine un mois avant sa mort. Je veux saluer sa soeur, son frère et sa famille, qui comptaient beaucoup pour lui. Il était heureux, bon vivant, souriant et surprenant. Un homme simple, bon, généreux, partageant ce qu'il aimait avec ceux qu'il aimait. Sa passion pour la pêche, vous l'avez rappelé, monsieur le président, l'a amené à découvrir tous les cours d'eau. Armé de patience, de mouches fabriquées maison, bien évidemment, de sa canne et de ses clopes roulées, il traquait la truite partout dans les ruisseaux de la Lozère.

Il n'y a aucune fatalité pour qui se bat pour une cause juste et noble. Il était l'homme du terroir, l'homme d'une région qu'il aimait plus que tout, mais aussi l'homme des idées de gauche qu'il ne lâcha jamais. Il savait écouter, respecter, discuter et débattre avec tous, sans distinction, parce qu'il aimait les gens, tout simplement. Alain Bertrand savait que, sans amour des gens, sans humilité et sans empathie, autrement dit sans humanité, il n'y a pas de vie politique digne.

La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion, présentée par le président du Sénat

mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du Sénat et de son président de créer, au sein de la Haute Assemblée, une commission d'enquête sur les politiques publiques menées durant la pandémie de covid-19 pour en tirer toutes les conclusions pour l'avenir de notre pays. Une telle commission d'enquête est indispensable pour comprendre les défaillances de notre système de santé, en particulier celles des missions des agences régionales de santé, mais aussi du pilotage national et de la gestion des stocks de médicaments et fournitures médicales. Notre objectif non pas de recopier le travail de nos collègues députés, mais d'y apporter un éclairage complémentaire sous le prisme de nos élus locaux qui ont été en première ligne durant la pandémie. Nous espérons que cette commission sénatoriale permettra de mettre en lumière un certain nombre de fragilités de notre système de santé dont l'origine remonte aux gouvernements précédents et actuel. La pandémie a apporté un terrible démenti aux politiques publiques qui ont oeuvré avec obstination à l'affaiblissement de notre système de santé et des infrastructures publiques de soin. Elle a mis à mal notre souveraineté sanitaire, comme le révèlent de manière dramatique les difficultés de notre industrie pharmaceutique à éviter les ruptures de stock de médicaments.

dont 1 milliard au détriment de l'hôpital public. En vingt ans, 100 000 lits ont disparu, dont 17 500 au cours des six dernières années. Notre objectif n'est pas de faire le bilan politique de l'action gouvernementale. Les élections sont et seront seules juges de l'action menée par l'exécutif : les résultats des municipales de dimanche semblent nous donner un aperçu de ce jugement. Sans esprit partisan, cette commission d'enquête permettra de faire la lumière sur les dysfonctionnements et leur origine, d'identifier les responsabilités et de mieux appréhender les moyens efficaces de lutte contre la pandémie qui nous frappe.

Monsieur le président, à mon tour, je veux vous remercier de l'initiative que vous avez prise en votre nom, mais aussi au nom de l'ensemble des présidents de groupe. Les commissions d'enquête - je parle sous le contrôle de M. le président de

Certes, nous avons dû affronter une très grave crise sanitaire ; certes, la covid-19 a tué, tue et tuera des centaines de milliers de personnes dans le monde. Mais ce virus, mes chers collègues, n'a pas ni conscience, ni projet d'envahissement, ni histoire, ni, du moins je l'espère, avenir. Ses seuls alliés potentiels sont les hommes et les femmes qui le diffusent auprès de la population. Monsieur le président, nous avons été frappés par une crise d'une violence inouïe.

n'aimerais pas être ministre dans de telles circonstances ! Le rôle du Sénat est de déceler ces failles et ces insuffisances pour les combler, les réparer et, surtout, les prévenir.

Certes, une deuxième vague réduirait à néant les efforts fournis jusqu'à présent et viendrait heurter de plein fouet un système de santé déjà très affaibli par la première vague. À cet égard, je vous invite à écouter ce que nous disent les soignants qui sont dans la rue, à Paris, aujourd'hui.

audit de l'État, préparation de la France à la gestion de la crise sanitaire et esquisse des perspectives pour la suite, soit autant d'étapes nécessaires, car nos concitoyens ont le droit et même le devoir de savoir. Cet esprit animera notre présence au sein de la commission d'enquête.

vote. Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons s'inscrit dans le cadre de l'exercice par le Sénat de ses missions de contrôle de l'action du Gouvernement prévues par la Constitution.

L'esprit à la fois critique et constructif de cette commission d'enquête nous permettra d'établir, du moins je l'espère, un bilan de l'action publique de ces derniers mois, qui n'ont ressemblé à aucun autre. Nous Nous accorderons une attention toute particulière à la cohérence et à la clarté de la communication de crise, à la gestion des fausses informations dans un contexte de grandes incertitudes et à l'analyse de l'éthique des décisions. Seront mises au clair les raisons du manque de masques, les décisions relatives aux durées de confinement et à ses modalités, ainsi que les conséquences de l'épidémie sur la continuité des soins. En tant que membre du groupe Les Indépendants, à l'origine de la mission d'information sur les pénuries de médicaments et de vaccins, j'accorderai une attention particulière au problème de la dépendance de la France à l'égard de la Chine en matière de produits de santé prioritaires, dans le prolongement du rapport de Jean-Pierre Decool, qui avait prédit ce danger dès le mois d'octobre 2018. Cette commission sera avant tout un exercice pragmatique, qui servira à alimenter l'action future en matière de santé publique. En accordant une large part au débat contradictoire, elle complétera et approfondira utilement l'exercice réalisé par l'Assemblée nationale. La France a trop longtemps négligé sa politique de prévention. Cet exercice de rigueur et d'humilité permettra à notre société d'avancer dans le bon sens.

mes chers collègues, dans ce contexte anxiogène, permettez-moi tout d'abord de saluer les professionnels, mais aussi les citoyens, nombreux à s'être investis par solidarité et responsabilité dans cette crise que personne n'avait prévue. Mes pensées vont vers ceux- résidents d'Ehpad, familles, soignants -qui ont vécu des drames familiaux et des décès brutaux, dans des circonstances plus que particulières. La crise sanitaire actuelle est inédite par son ampleur. Elle a touché le monde entier et percuté tous les pans de la société. Il est donc logique que les institutions évaluent les politiques publiques à l'oeuvre, mais également s'interrogent sur la gestion par les pouvoirs publics de cette crise. L'exigence de transparence est légitime pour discerner ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné et ce qui doit être amélioré. C'est dans cet esprit que la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui a entamé ses travaux en avril, s'est dotée des pouvoirs d'enquête dès le 16 juin dernier. En parallèle, le Président de la République a installé, le jeudi 25 juin, la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise du covid-19 et l'anticipation des risques pandémiques. Je souhaite insister sur un point : cette mission n'empiétera pas sur les prérogatives du Parlement. Il s'agit d'un travail complémentaire des travaux des assemblées, multidisciplinaire, mené par des experts des champs scientifique, économique, administratif et sociétal. La mission rendra un rapport en fin d'année ; un rapport d'étape est prévu à l'automne. Au regard de l'ampleur de la crise, il est opportun que chaque institution se dote d'outils appropriés pour évaluer la gestion de celle-ci et ainsi mieux anticiper les crises futures. Par ailleurs, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a ouvert lundi 8 juin une vaste enquête préliminaire sur la gestion de la crise en France. Si nous avons entendu des propos, sur certaines travées,

Pour autant, la situation ne saurait être exploitée à des fins politiciennes. Nous voulons une analyse approfondie, lucide, rigoureuse, objective, totalement transparente, une analyse à laquelle nous procéderons, pour ce qui nous concerne, avec humilité, mais sans céder à des penchants politiciens. Mes chers collègues, soyez rassurés, il n'y aura de notre part aucune complaisance à l'égard des choix faits par le Gouvernement avant et durant la crise sanitaire. Cependant, les décisions prises devront être évaluées au regard des connaissances et du consensus scientifique du moment. Veuillez conclure, ma chère collègue. Aussi, notre groupe est résolument favorable à toute initiative visant à comprendre, à prévenir et à améliorer la gestion des crises sanitaires,

Nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution présentée par M. Gérard Larcher, président du Sénat, tendant à créer une commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion.

Des sujets délicats devront être soulevés avec la plus grande prudence, mais également avec la plus grande détermination pour mettre en lumière ce qui a bien fonctionné, relever les initiatives locales qui pourraient être généralisées, mais aussi nos défaillances techniques et organisationnelles ou bien les potentiels conflits d'intérêts ayant pu déboucher, même indirectement, à des prises de décisions ni totalement libres ni totalement éclairées. M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, le rappelait : sa génération aura connu le chômage de masse, la transition écologique, le sida et la covid-19. Au moment du dépôt de ce texte, et depuis le 31 décembre dernier, cette crise a emporté la vie de 433 259 personnes à travers le monde, dont 29 436 en France. La détermination de nos soignants et leur engagement sans faille dans un contexte de relative ignorance du mal qu'ils devaient combattre aux côtés des malades les ont plongés dans de nombreuses semaines de dévouement total, tout en les isolant de leurs proches. Les applaudissements quotidiens à vingt heures constituaient la reconnaissance des Français envers celles et ceux qui travaillaient sans relâche. Le Ségur de la santé apportera des réponses pour revaloriser leurs professions. Aussi, il était du devoir des parlementaires de constituer à l'Assemblée nationale et ici, au Sénat, des commissions d'enquête, afin de tirer le bilan de cette crise, pour proposer ensuite des améliorations et des garanties pour une meilleure efficacité de notre système. Ainsi, celui-ci sera plus réactif et adaptable aux crises sanitaires majeures. Il s'agit enfin de lui donner la capacité de prendre avec assurance des décisions libres, éclairées, justes et les plus efficientes possible. C'est pourquoi, mes chers collègues, les membres du groupe Union Centriste voteront unanimement en faveur de cette proposition de résolution.

par les grandes épidémies. Nous nous sommes crus à l'abri, sans doute parce que nous avons été habitués aux progrès de la science, qui repousse toujours les limites de la maladie, comme aux bienfaits de l'État-providence et de son administration protectrice. Si cette crise est exceptionnelle, elle n'était pas non plus totalement imprévisible. Bien sûr, son ampleur a rendu nécessaire la prise de décisions très complexes, dans un temps extrêmement bref. Nul ne contestera dans cet hémicycle la difficulté d'agir dans de telles circonstances, y compris en créant en quelques jours un régime juridique dérogatoire au droit commun. Toutefois, sur le temps long, et sans faire affront au travail admirable des personnels soignants, la crise a été le révélateur des profonds dysfonctionnements de notre système de santé, qui se sont sédimentés au fil des gouvernements successifs. Je pense ainsi à la lourdeur des circuits administratifs, à la situation des Ehpad,

de responsabilité et de défense de l'intérêt général que le groupe du RDSE soutiendra unanimement la création de cette commission d'enquête. Personne ne demande

la commission d'enquête chargée d'évaluer la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, sur les conclusions de son rapport. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

il me revient la mission d'ouvrir notre débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La multitude des problématiques posées par cet accident

Le 26 septembre dernier, au coeur d'une métropole, cet accident a provoqué la dispersion dans l'environnement de nombreux produits chimiques, dont le nombre et les effets demeurent encore, pour une large part, inconnus.

et celles qui entourent le sujet délicat du suivi sanitaire des populations exposées. Avoir su éviter une catastrophe ne doit pas nous faire oublier les lacunes opérationnelles importantes dont souffre le pilotage local et central des catastrophes sanitaires.

La réponse globale apportée sur le terrain, sous l'égide du préfet de département, a permis d'éviter une catastrophe. Pour autant, les interventions sporadiques et non coordonnées de plusieurs ministres, chacun dans leur secteur de compétences, ont pu donner l'impression d'une certaine cacophonie et, peut-être, d'un opportunisme purement politique. Ainsi le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a-t-il décidé de lever la consigne sur les produits laitiers plusieurs jours avant que l'expert sanitaire rende publics les résultats des analyses des produits agricoles. Comment voulez-vous que la population s'y retrouve ? Plus préoccupants ont été nos constats sur le suivi sanitaire des populations exposées au nuage de fumée. L'épidémie de covid-19 a contraint les décideurs publics à tenir compte de l'incertain dans la protection des populations d'un danger sanitaire. C'est exactement l'enseignement que nous tirons, Nicole Bonnefoy et moi-même, de l'analyse de la gestion de crise de l'accident de

Effectivement, sans attendre qu'un danger soit strictement identifié, plusieurs risques nous paraissent justifier un suivi sanitaire d'envergure. Tout d'abord, je pense aux lacunes persistantes des analyses réalisées sur les prélèvements d'air. Les décideurs publics semblent s'être un peu vite satisfaits de résultats partiels, alors que des incertitudes demeurent sur le délai de diffusion des dioxines et des furanes dans les sols ou sur les conséquences à plus long terme de certains composés du phosphore. se pose la question des effets cocktails des molécules contenues dans le panache de fumée, dont les interactions peuvent produire dans l'organisme humain des effets largement méconnus. il y a la question controversée de la dispersion de particules d'amiante au moment de l'explosion du toit des entrepôts abritant les produits stockés. Il nous paraît donc évident qu'à l'égard de certains risques ciblés l'inapplication d'un principe de précaution en matière de suivi sanitaire, au motif d'une absence de certitude scientifique, ne peut plus se justifier. C'est pourquoi, outre la consécration d'un tel principe au rang législatif, nous recommandons que soient ouverts deux registres de morbidité, relatifs l'un aux cancers généraux et l'autre aux malformations congénitales. Je serais heureuse, madame la secrétaire d'État, de recueillir votre sentiment sur ce point. S'il est une leçon que les événements récents, à défaut de ceux qui sont plus anciens, doivent désormais nous inspirer,

à l'issue de huit mois de travaux quelque peu perturbés par la crise sanitaire, nous avons formulé une quarantaine de recommandations s'inscrivant dans six axes principaux, afin d'améliorer la prévention et la gestion des accidents industriels majeurs. la secrétaire d'État, que vous preniez ce rapport pour ce qu'il est, soit un outil destiné à éviter qu'une telle situation ne se reproduise, et non une dénonciation de votre politique, comme j'ai pu l'entendre ou le lire dans la presse. Avant toute chose, nos travaux ont mis en évidence des angles morts importants dans la politique de prévention des risques, en particulier la difficulté de l'administration à accéder en temps réel à l'information relative à la localisation et à la composition des produits stockés dans un site Seveso. Le nombre réduit de sanctions prononcées à l'encontre des industriels après le constat de manquements aux obligations légales et réglementaires semble relever d'une certaine passivité en matière de contrôles, notamment pour ce qui concerne le risque incendie, première source d'accident industriel. Ensuite, nous avons constaté que le public est le grand absent de la politique de prévention des risques : 90 % des Français se sentent mal informés sur les risques industriels et technologiques et 10 % à peine affirment savoir comment réagir en cas d'accident. Les élus et les associations de protection de l'environnement ont également formulé des critiques sur le fonctionnement des instances de concertation. L'accident de l'usine Lubrizol révèle révèle donc, une fois encore, un manque de culture du risque et de la sécurité. Pour tenir compte de ces fragilités, ma collègue rapporteure et moi-même demandons notamment l'augmentation de la fréquence des exercices, la diversification de la composition des structures de concertation, le renforcement des obligations des exploitants en matière de prévention du risque incendie et le développement des mutualisations entre opérateurs à l'échelle d'un bassin de risque. Plusieurs des mesures que vous avez soumises à consultation vendredi dernier, madame la ministre, reprennent ces recommandations, au moins pour partie. C'est une bonne chose.

pour renforcer l'information des élus sur les risques industriels, mais aussi sur les risques sanitaires et sur les risques climatiques. J'espère, madame la ministre, que vous pourrez contribuer à cette action qui nous semble tout à fait essentielle. En matière financière, nous proposons de proroger le crédit d'impôt en faveur des ménages qui réalisent des travaux dans leur logement en lien avec un PPRT, mais aussi d'instituer une avance aux particuliers, car beaucoup d'entre eux ne paient pas d'impôt sur le revenu. Nous avons aussi affirmé la nécessité que les victimes de l'accident ne subissent aucune franchise. Cette mesure est tout sauf symbolique pour les personnes modestes touchées par l'incendie. Je conclurai mon propos en vous interrogeant sur deux points, madame la ministre.

alors que le nombre de contrôles, lui, a été divisé par deux. Vous pouvez évidemment compter sur notre soutien s'il s'agit d'engager le combat contre Bercy pour atteindre cet objectif. Surtout, comment comptez-vous mieux associer les citoyens à la politique de prévention des risques et renforcer l'information du public, en particulier les riverains des sites classés ? La parole

je souhaite d'abord vous remercier de me donner de nouveau l'occasion d'échanger avec vous sur les suites de l'accident industriel de Lubrizol. Je veux rappeler, à titre d'introduction, que le Gouvernement a fait face aux conséquences environnementales de cet accident avec une parfaite transparence. L'analyse complète de l'état des milieux du département de Seine-Maritime, fondée sur des prélèvements dans les 112 communes exposées aux retombées de suie, a été présentée au comité pour la transparence

Des résultats complémentaires sont encore attendus pour les zones plus éloignées de l'incendie, dans l'Oise et le Nord. Je le souligne, c'est la première fois qu'un protocole de surveillance aussi ambitieux est mis en oeuvre.

si un accident industriel survient, la liste des produits concernés par l'incendie et des substances susceptibles d'être émises du fait de celui-ci sera désormais mise à disposition du public. Par ailleurs, l'analyse des causes du développement rapide de l'incendie nous conduit à revoir les mesures de compartimentage, la disposition des stockages de produits et la conception des cuvettes de rétention. Pour que les industriels soient mieux préparés à la gestion d'un accident, l'obligation de réaliser un plan d'opération interne, c'est-à-dire un plan de gestion de crise interne à l'établissement, sera désormais étendue à l'ensemble des sites Seveso. La mise en oeuvre de ces plans d'urgence devra être testée lors d'exercices réguliers : tous les ans pour les sites Seveso seuil haut ; tous les trois ans pour les autres installations. Les principaux textes d'application de ce plan d'action sont soumis à la consultation du public depuis vendredi dernier, et les autres le seront d'ici à la fin de l'été. Je me suis engagée à renforcer les contrôles une augmentation de 50 % du nombre d'inspections d'ici à la fin du quinquennat. Après avoir fait le bilan des possibilités d'allégements de tâches administratives,

Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale m'a été remis, et je souhaite que ses propositions viennent enrichir le plan d'action du Gouvernement. Pour ce qui concerne les PPRT, je peux vous confirmer que 385 plans sur 390

votre rapport, la nécessité de créer une véritable culture du risque industriel. On le sait, de nombreux dispositifs réglementaires visent à associer les élus et à informer les citoyens et les entreprises

Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions ; je laisse la parole à Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, sur les sujets

l'incendie de l'usine Lubrizol, site classé Seveso seuil haut, survenu dans la nuit du jeudi 26 septembre dernier, a suscité une profonde inquiétude dans l'ensemble de la population rouennaise et, plus largement, chez nos concitoyens concernés par les conséquences du panache de fumée, et soulevé de nombreuses interrogations légitimes sur les effets sur la santé de cet incident industriel grave.

populations. Je souhaite en particulier rappeler la qualité et la diligence du système de soins et des autres services de l'État, ainsi que des expertises mobilisées.

notamment par l'édiction de recommandations sanitaires, et à surveiller les effets sanitaires immédiats, afin de déterminer les prises en charge adaptées et d'ajuster l'offre de soins si la situation l'exigeait. Aucun cas grave n'a été rapporté durant cette phase aiguë, dont le bilan sanitaire a été confirmé par l'Agence Afin d'assurer une surveillance de la population dans les jours suivant l'incendie, Santé publique France a été saisie par le ministère des solidarités et de la santé pour la réalisation en urgence d'une synthèse concernant l'incidence sanitaire observée. Une surveillance renforcée de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine a été mise en oeuvre par l'ARS Normandie, qui a effectué des analyses tout de suite après l'incendie, en complément des analyses régulières du contrôle sanitaire des eaux. Le ministère a suivi avec attention les résultats des analyses réalisées par les différents services de l'État pour caractériser la contamination dans les autres milieux, concernant notamment plusieurs substances préoccupantes, afin, le cas échéant, d'adapter les recommandations sanitaires diffusées auprès des populations. n'a pas été nécessaire. En effet, les analyses n'ont mis en évidence aucun résultat non conforme aux valeurs seuil. Le ministère des solidarités et de la santé a par ailleurs procédé à l'évaluation précise des conséquences de l'incendie

La commission d'enquête a formulé plusieurs recommandations ; sept d'entre elles relèvent du champ du ministère des solidarités et de la santé. Nous aurons probablement l'occasion d'échanger, au cours de ce débat, Nous partageons évidemment l'objectif qui consiste à améliorer la capacité à protéger les populations. Deux questions m'ont été posées. Pour ce qui concerne la création de registres de morbidité, la mise en place de nouveaux registres ne nous semble pas opportune compte tenu du périmètre couvert par les registres existants. Néanmoins, des améliorations sont toujours possibles. S'agissant des cancers, nous étudions la possibilité d'estimer leur incidence à l'échelon infradépartemental, ce qui répondrait à la préoccupation

Concernant enfin le suivi sanitaire renforcé, nous vous rejoignons évidemment sur la nécessité de disposer d'un suivi à moyen et à long terme des conséquences sanitaires de l'incendie ; quatre approches ont été identifiées à cet effet par Santé publique France. Nous allons maintenant

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Or le rapport relève très justement que le principe de précaution aurait dû prévaloir dès le départ, qu'il devrait guider le suivi sanitaire de la population et des salariés sur le long terme, l'ouverture de registres de morbidité étant

un dispositif législatif autorisant le déclenchement immédiat, après ce type d'accident, d'enquêtes sanitaires et environnementales

d'une meilleure association des élus locaux, en particulier des maires, dans la gestion de crise, dans le contrôle des sites, dans les exercices de sécurité civile. Il est indispensable que l'État considère enfin les élus locaux comme des partenaires à part entière. Quelles consignes entendez-vous donner en ce sens ? La parole

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de saluer le caractère complet de ce rapport à l'occasion de son adoption par la commission d'enquête. qu'il contient devront bien sûr être prises en compte. Je souhaite, mesdames les ministres, attirer votre attention sur l'importance du rôle de l'information, soulevée par ce rapport, et qui me semble primordiale. La gestion d'une crise de l'ampleur de celle de l'incendie de l'usine Lubrizol

Est-on sûr, aujourd'hui, qu'un véritable suivi épidémiologique sérieux a bien été mis en place ? Des prélèvements de carottes ont-ils été effectués ? S'agissant de la réparation des préjudices, si la première phase s'est déroulée à peu près convenablement, cela ne semble pas être le cas de la deuxième phase : la paperasse a pris le dessus sur la fluidité.

Je précise également que l'Ineris met à disposition une cellule d'appui aux situations d'urgence qui permet de modéliser le panache d'un incendie dans les meilleurs délais. En l'occurrence, dans le cas de l'accident de l'usine

Je peux vous assurer également que les prélèvements conservatoires, c'est-à-dire portant sur l'eau potable et sur la chaîne alimentaire, et les prélèvements environnementaux ont été effectués dans l'ensemble des communes susceptibles d'avoir été affectées par le panache, indépendamment des limites administratives. Aujourd'hui, nous avons pu exploiter tous les prélèvements de Seine-Maritime ; dans le courant du mois de juillet, nous disposerons des prélèvements

le 26 septembre 2019, quand l'incendie hors norme de l'usine Lubrizol s'est déclaré, j'étais sur place en tant que président du conseil départemental de la Seine-Maritime, fonction que j'occupais à l'époque. Je peux témoigner à la fois de la violence du choc et du caractère exemplaire des premières réactions. L'engagement des salariés de l'usine a été sans faille. Il a été immédiatement relayé par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, puis par les services homologues de six départements voisins. C'est sans doute grâce à cet engagement que le sinistre n'a fait ni morts ni blessés et n'a endommagé aucune habitation. Pour autant, l'accident a révélé un certain nombre de faiblesses dans notre système de prévention et de prise en charge des accidents industriels. La prévention est l'un des enjeux majeurs que font ressortir les conclusions de notre commission d'enquête, dont je salue au passage l'excellence du travail.

Pour que cette réaction soit optimale, il faut que toutes les autorités appelées à intervenir soient parfaitement coordonnées, en particulier la préfecture et les élus. Or tel n'est pas le cas. Le plan communal de sauvegarde élaboré par le maire n'est pas articulé avec le plan particulier d'intervention du préfet. Les élus locaux ne sont pas systématiquement associés aux exercices de sécurité,

crée la confusion dans l'esprit des administrés, lesquels, spontanément, s'adressent à leur maire dans l'urgence. Madame la ministre, comment comptez-vous assurer l'articulation entre le préfet et le maire en cas de sinistre majeur,

De fait, elles sont associées aux différentes étapes clés de la vie d'un site industriel. Je rappelle que les élus sont associés dès la phase d'autorisation d'une installation industrielle : l'étude de dangers et l'étude d'impact sont réalisées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation. Une enquête publique est organisée, organisée, et tous ces documents sont alors mis à disposition du public. En parallèle, un avis spécifique est demandé aux collectivités territoriales et à leurs groupements directement concernés par le projet. Les élus sont aussi associés dans les instances de suivi de la vie d'une installation industrielle ; ils participent notamment aux commissions de suivi de site (CSS), qui sont obligatoires autour des sites Seveso seuil Ils sont également représentés dans les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels, qui sont les structures de concertation locales autour des grandes plateformes industrielles. Les collectivités déclinent les dispositifs réglementaires visant à garantir la diffusion de la culture du risque sur leur territoire ; vous savez que le document départemental sur les risques majeurs est mis à disposition des élus par les préfectures ; c'est sur cette base que les élus élaborent les documents d'information communaux sur les risques majeurs. pour ma part, qu'il faut aller plus loin ; tout l'objet de la mission sur la modernisation de la culture du risque que je souhaite lancer à la rentrée sera là. On voit bien en effet qu'en définitive, malgré ces dispositifs d'information des élus, malgré les enquêtes publiques, malgré l'existence des commissions de suivi autour des sites industriels, industriels, la culture du risque n'est pas suffisante dans notre pays. Il s'agit donc de renouveler cette culture, de faire plus participer les citoyens, d'associer davantage les collectivités, par exemple lors des

faut, me semble-t-il, aller plus loin encore pour tirer les conséquences de cette recommandation. Dans les faits, depuis 2009, on constate de multiples reculs et une instabilité du droit de l'environnement, constat partagé par nombre de juristes de l'environnement et responsables d'ONG. Au prétexte d'une simplification, droit ne cesse de se complexifier, avec pour corollaire un affaiblissement de l'efficacité des normes et de la démocratie environnementale, mais aussi une insécurité juridique pour les porteurs de projets. On peut notamment citer la création du régime de l'enregistrement, les relèvements de seuils, les dispenses d'évaluation environnementale des projets au cas par cas, les suppressions de consultations obligatoires. Cette régression du droit de l'environnement est aggravée par la chute

et en se donnant les moyens d'appliquer le droit, une justice spécialisée. Aussi, madame la ministre, le Gouvernement prévoit-il de renforcer l'efficacité du droit de l'environnement et de mettre en oeuvre une politique de sanction réellement dissuasive ? La parole

confondre la simplification des démarches avec le degré de protection apporté. Vous avez raison de souligner que les gouvernements successifs, depuis une dizaine d'années, ont essayé de simplifier les procédures,

vendredi dernier, vise à renforcer la transparence sur les accidents et leurs conséquences, à prendre des dispositions supplémentaires pour empêcher la survenue de nouveaux incendies d'ampleur et à accroître les moyens de contrôle- j'ai eu l'occasion d'évoquer S'agissant des sanctions, je partage tout à fait l'idée qu'il faut s'assurer que les poursuites pénales ont bien lieu et que les sanctions sont réellement dissuasives. C'est bien tout le travail que nous avons engagé avec Mme la garde des sceaux, Nicole Belloubet,

remercie, madame la ministre, de votre réponse. Dans l'actualité de cette semaine, la Convention citoyenne pour le climat a montré une attente forte des citoyens, de juger sévèrement les atteintes à l'environnement la création d'un crime d'écocide. Il s'agit d'une idée majeure. Sans trancher ici le débat de savoir si ce crime devrait être reconnu dans notre droit national ou à l'échelon international, cette proposition appelle à un véritable renforcement du droit pénal environnemental, qui prendrait

Sénatrice de la Gironde, je rappelle que sur les 1 312 installations classées Seveso en France, 157 se situent en Nouvelle-Aquitaine. Et mon département est celui qui en compte le plus. Lors de votre audition, madame la ministre, j'avais abordé la problématique de la culture du risque en France, en lien avec les différentes visites que j'ai effectuées dans mon département où sont implantés 35 sites Seveso+, ainsi que le besoin des maires d'être accompagnés, notamment pour ce qui concerne la sensibilisation de leurs concitoyens. En fin d'année dernière, lors de son audition, le président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs avait attiré notre attention sur l'importance d'une information plus transparente, mieux partagée entre les services de l'État, les entreprises concernées et les élus locaux.

Un chiffre est avancé dans le rapport : 90 % des Français se sentent mal informés sur les risques que présentent les installations industrielles et chimiques. Si notre pays est doté d'outils et de structures garantissant l'information et la participation du public, la question de la composition de ces structures a été posée- c'est un élément du rapport -, de même que le type de système d'alerte utilisé. De façon transversale, c'est la question de la coordination des et des collectivités territoriales dans la réponse opérationnelle à apporter dans l'urgence ... Il faut conclure ! ... et pour renforcer l'appropriation de la gestion des risques industriels

au document départemental sur les risques majeurs. Néanmoins, ces dispositifs paraissent aujourd'hui très formels et ne permettent pas d'assurer une sensibilisation large, efficace et pédagogique de la population face aux risques industriels. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une mission pluridisciplinaire pour renforcer la culture du risque. Il s'agira, notamment, de poser un diagnostic partagé avec les parties prenantes pour redéfinir les enjeux et les attentes en matière d'information et d'acculturation au risque, d'examiner la pertinence des dispositifs existants et d'identifier les outils et les canaux les plus efficaces pour sensibiliser le grand public avec pédagogie. Il s'agira aussi de proposer des pistes d'approches participatives mobilisatrices pour mieux associer les élus. Vous savez que la France est dotée d'un réseau national d'alerte composé d'environ 4 500 sirènes, sous le pilotage du ministère de l'intérieur. Ces sirènes sont testées le premier mercredi du mois dans les plus grandes villes. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont aussi largement utilisés par les préfectures, ce qui peut améliorer l'information. Par ailleurs, d'autres dispositifs sont à l'étude par le ministère de l'intérieur, notamment pour faire sonner les téléphones portables dans les zones en cause. Il existe au demeurant une directive européenne de 2018 qui prévoit que les alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communication. Le Gouvernement se prépare à mettre en oeuvre cette directive.

des ateliers d'écriture en invitant les acteurs du territoire compétents à travailler ensemble pour que les informations transmises en cas d'incident industriel puissent être comprises et assimilées par les populations. Ce travail d'écriture n'a jamais eu lieu et les mêmes erreurs de communication sur la qualité de l'état sanitaire de l'air ont été reproduites en 2019. Elles ont largement contribué à discréditer la parole des autorités, car celles-ci n'étaient pas « entendables Pensons simplement à la cacophonie qui a régné après la survenance de l'incident, avec six déplacements ministériels en une semaine pour autant de déclarations divergentes Que comprend le public lorsqu'on lui dit qu'il n'y a pas de toxicité alors même qu'il voit un incendie hors norme dégageant un impressionnant panache noir ? Que comprend le public quand le préfet parle d'une qualité de l'air « habituelle » alors qu'il est, dans le même temps, soumis à des effluves extrêmement malodorants, qu'il ressent des irritations, des nausées et des maux de tête ? Face aux crises, l'État ne peut pas avoir raison tout seul, notamment parce que ces crises sont complexes et que l'État central ne saurait, par nature, avoir une complète connaissance du terrain, au contraire des associations et des collectivités. Nous avons besoin de cette subsidiarité. La France dispose d'associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui exercent une mission de service public aux côtés de l'État, et leur caractère professionnel est avéré. Pourquoi laisser de côté la parole de ces associations expertes ? Madame la ministre,

association a décidé de suspendre la diffusion de son indice qui, de fait, cible des polluants comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules PM10 et l'ozone, qui ne sont pas réellement représentatifs des substances émises pendant l'incendie.

important à jouer dans la mise en place de mesures spécifiques de prélèvements de l'air à la suite d'un incendie. Vous savez que les exploitants de sites Seveso, qui ont un plan d'opération interne, seront appelés à identifier

2019, les riverains de l'usine Lubrizol, à Petit-Quevilly, sont réveillés, le 26 septembre vers trois heures du matin, par des explosions, bien avant les premières alertes officielles, et sortent dans la rue, inquiets, s'exposant directement aux fumées et aux produits toxiques. Enfin informée, Mme la maire de Petit-Quevilly déclenche le système d'alerte à six Mais les populations et les élus des autres communes affectées, de la rive gauche comme de la rive droite, devront encore attendre. Ce n'est qu'à sept heures quarante-cinq que la préfecture déclenchera les sirènes d'alerte pour les informer. De nombreux élus vont protester contre ce traitement inadapté de l'information par les services de l'État. d'enquête pointe du doigt une réelle défaillance de communication de la part de ces derniers dans la gestion de cette crise. À vouloir éviter la panique, ils ont créé un vide propice à l'inquiétude et à l'angoisse. De plus, la sous-exploitation des réseaux sociaux par ces mêmes services n'a pas permis de diffuser des explications sur le déroulement des événements ni d'informer les populations sur les conduites à tenir. Contrairement à d'autres préfectures, celle de Seine-Maritime n'a pas signé de convention qui lui aurait permis d'analyser la crise médiatique et de détecter, en amont, les activités sur les réseaux sociaux, pour mieux les maîtriser. Or, au cours d'une visite par la commission dans la vallée de la chimie, à Lyon, nous avons constaté qu'il est possible aux grands acteurs, publics et privés, de travailler en concertation sur les stratégies de communication de crise. Ne faudrait-il pas faire de cette initiative une règle sur notre territoire ? Chez nous, le 26 septembre, il fut bien difficile de faire la part des choses entre mesures de mise à l'abri, de confinement, voire absence totale de consignes. Madame la ministre, vous avez mentionné le système d'alerte du et vous avez annoncé qu'il serait mis en place en 2021.

dont je rappelle qu'elle ne relève pas directement de mon ministère, s'imposait. Il est donc en cours pour clarifier et moderniser la doctrine de communication de l'État, à l'échelle centrale comme à l'échelle locale. Il s'agit aussi d'avoir un meilleur suivi de l'activité des réseaux sociaux de façon à identifier très en amont les attentes du public et de prévenir, le cas échéant, la diffusion de fausses nouvelles.

faire sortir de chez eux les riverains la nuit en déclenchant la sirène avant d'avoir mis en place les moyens permettant de maîtriser l'incendie.

cette enceinte, élue directement de ces territoires, présente dans les heures et jours qui ont suivi l'incendie, je peux porter témoignage, comme je l'ai fait dès le lendemain en posant une question d'actualité au Gouvernement, de la gestion de cette crise

Est-il normal que ce soient les gendarmes qui soient venus informer les maires pour leur demander s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange dans leur commune ? Dès lors, comment les élus peuvent-ils répondre aux inquiétudes de leurs administrés ?

Autre problème, selon la commission d'enquête, « 62 % des élus font part d'un manque d'information sur les risques industriels et 78 % sont peu ou pas associés aux exercices de sécurité civile

Alors que vont s'installer les nouvelles intercommunalités, êtes-vous prête à accompagner les élus, humainement et financièrement, dans des zones à risque telles que les nôtres pour l'élaboration

dans les commissions de suivi de site et dans les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels. Ils ont également communication du document départemental sur les risques majeurs, document sur la base duquel ils

M. René Danesi. Madame la ministre, l'excellent rapport de la commission d'enquête relève que notre organisation de la gestion de crise est inadaptée aux risques industriels et technologiques majeurs.

les dirigeants de Lubrizol étaient alertés depuis 2014 par les rapports de risques établis annuellement par leur assureur, FM Global, sur les failles de leur dispositif anti-incendie. Mais ils n'ont pas estimé utile de réagir, car selon eux « les équipements de Rouen étaient, au jour de l'incendie, conformes à la réglementation en vigueur Le rapport du Sénat souligne non seulement l'insuffisance des contrôles de l'administration, mais aussi la mauvaise information des pouvoirs publics par certaines entreprises. Ainsi, l'administration n'avait pas connaissance de tous les produits stockés ni de leur quantité. Certes, Certes, l'instruction du Gouvernement du 31 décembre 2019 recommande « de confronter les éléments présentés par l'exploitant dans des documents, comme les études de dangers, avec la réalité du terrain ». Certes, le rapport sénatorial suggère prudemment d'établir « d'éventuelles passerelles entre l'administration et les assureurs, au-delà de la synthèse réalisée par l'exploitant ».

les exploitants d'usines de type Seveso haut à communiquer immédiatement à l'administration compétente les rapports complets de leurs assureurs

toutes deux un objectif commun : prévenir les accidents de grande ampleur. Du côté des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement, il s'agit de prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement, alors que pour les assurances, les assurances, il s'agit davantage de prévenir les dommages économiques graves à l'outil de travail et au stock de valeurs, comme les produits finis. La mission d'information de l'Assemblée nationale nous avait recommandé d'imposer aux exploitants des sites Seveso de mettre à la disposition du service des installations classées les rapports de visite des experts d'assurance. Nous avons engagé des concertations avec les assureurs et les fédérations professionnelles pour y travailler. Dans le cadre des arrêtés soumis à consultation, il est prévu d'imposer aux exploitants d'entrepôts ou de sites Seveso de mettre à disposition

Néanmoins, elles ne sont pas toujours reconnues à leur juste place par les services déconcentrés de l'État. Sur ce point, notre rapport appelle à un changement de regard de la part de ces services.

L'ensemble de la commission a insisté sur la nécessité d'une formation permanente des citoyens pour mieux les sensibiliser aux risques. Cela passe aussi par des exercices inopinés, qui ne sont pas sans conséquence puisqu'ils perturbent la vie quotidienne de nos concitoyens. Madame la ministre, comment le Gouvernement peut-il favoriser l'organisation des exercices grandeur nature, dans un esprit de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire ? Seriez-vous favorable à la création d'un fonds dédié aux coûts des exercices inopinés ? La parole est à Mme la ministre.

aux différentes étapes de la vie d'un site industriel. De fait, comme je l'ai souligné, les élus sont associés à la procédure dès l'autorisation d'une installation industrielle. Les études de danger et l'étude d'impact, qui sont systématiquement réalisées dans le cadre du du dossier de demande d'autorisation, font ensuite l'objet d'une enquête publique, ce qui permet de porter ces informations à la connaissance du public. En parallèle de l'enquête publique, un avis spécifique est demandé aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont directement concernés par le projet.

pour la prévention des pollutions et des risques industriels, qui organisent des concertations locales autour des grandes plateformes industrielles. Par ailleurs, les collectivités territoriales déclinent les dispositifs réglementaires pour garantir la diffusion de la culture du risque sur leur territoire. À l'échelle des départements, les préfets élaborent un document départemental sur les risques majeurs, qui est mis à disposition des élus. Sur cette base, les élus rédigent leur document d'information communal sur les risques majeurs, le Dicrim. Dans le cadre de la mission sur la culture du risque que je lancerai à la rentrée, je souhaite que le rôle des élus dans l'élaboration d'une culture du risque soit renforcé. On pourrait peut-être organiser une journée nationale dédiée à la prévention des risques,

dans la gestion des risques. Je pense, notamment, à l'élaboration des plans communaux de sauvegarde grâce auxquels les collectivités se préparent en cas de survenance d'un risque technologique ou naturel.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, l'incendie de l'usine Lubrizol a remis sur le devant de la scène les dangers potentiels de certaines activités industrielles. À l'heure où l'on prône légitimement la réindustrialisation stratégique de la France, il ne faudrait pas que ce genre de catastrophe entraîne la délocalisation de ces industries. Dans le cas d'activités impliquant des matières dangereuses, il faut donc des standards élevés de sûreté. C'est pourquoi l'État doit assurer le contrôle et être le garant du respect des standards auprès des grandes et surtout des petites entreprises. La France dispose d'entreprises industrielles performantes, formées techniquement, soumises à des réglementations exigeantes, comme le classement Seveso seuil haut. Faisons confiance à ces professionnels ! Il faut également un contrôle de l'application des réglementations. Plus c'est technique et dangereux, plus il faut contrôler. L'incendie de l'usine Lubrizol a révélé aussi la nécessité d'une meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales. Aux côtés des services de l'État, les collectivités territoriales ont de nombreuses responsabilités en matière de risques industriels : sensibilisation du public, délivrance des autorisations d'urbanisme, participation à la gestion de crise, assistance et information des citoyens en cas d'accident. Mais les élus locaux, en première ligne lors d'une catastrophe de grande ampleur, ne disposent pas toujours des moyens et des informations nécessaires. Or ils doivent répondre aux besoins et aux inquiétudes de la population. La commission d'enquête a formulé plusieurs recommandations pour assurer une meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales. Il faudra notamment renforcer l'articulation entre plan particulier d'intervention (PPI) et plan communal de sauvegarde (PCS) pour améliorer la réponse opérationnelle et renforcer l'appropriation de la gestion des risques industriels et technologiques par les élus. Madame la ministre, il faut faire confiance aux élus locaux, car ce sont eux qui ont la confiance des habitants. Quel est votre avis sur cette recommandation ? La

essentiel à jouer dans la prévention des risques, y compris en cas de survenance d'une crise telle que l'incendie de Lubrizol. Les élus ont ainsi un rôle de premier plan à jouer pour informer et rassurer les populations.

Les éléments disponibles relatifs aux conséquences de l'accident sur l'eau, les sols, les milieux naturels et la biodiversité sont ainsi limités. Durant nos travaux, je me suis attaché à éclaircir la question de l'effet sur l'eau non seulement de l'incendie, mais également des procédés déployés pour l'extinction Lors de son audition au mois de novembre, le ministre de l'intérieur nous confirmait que la pollution de la Seine avait été inévitable, dans la mesure où les eaux d'extinction s'étaient tout d'abord écoulées par les sols. Selon lui, un système de sécurité aurait néanmoins été mis en oeuvre avant que des pollutions manifestes de la Seine aient lieu, par le confinement des eaux d'extinction dans un bassin, ou darse. Le 18 février dernier, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a rendu les résultats de sa campagne de suivi de la qualité des eaux de cette darse. Les analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de trace de pollution hors de la darse. En revanche, elles font ressortir que l'incendie a eu une incidence certaine sur la qualité des sédiments dans la zone de la darse.

installée non loin du fleuve Loire dans sa partie amont, je n'ose imaginer les conséquences pour tous les territoires situés en aval ! L'eau est notre patrimoine commun. Cette ressource indispensable à la vie est de plus en plus fragilisée par les activités humaines courantes. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, quelle réponse vous envisagez d'apporter à cette question essentielle de la préservation de l'eau en cas de catastrophe industrielle ? La parole est à Mme la ministre. Je veux vous

inspectés. Nous sommes particulièrement vigilants quant à la protection des cours d'eau. Les produits dangereux pour les milieux aquatiques sont ainsi pris en compte dans le classement sous le régime Seveso des sites industriels.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a créé, en quelques heures, un climat de panique bien compréhensible dans la ville et bien au-delà. Cette catastrophe, hormis le volet sanitaire, largement évoqué dans ce débat, a mis en avant un réel problème touchant notre dispositif de gestion et de communication en matière de crise lorsque survient un incident, en l'occurrence un incendie, dans un site industriel classé. La commission d'enquête, dont je salue le travail, a notamment mis en lumière le manque d'information des Français sur les risques que présentent les installations industrielles et chimiques situées à proximité de leur habitat, ainsi que sur la réaction à adopter en cas d'incendie de ce type.

Cette gestion hasardeuse de la communication de crise à l'heure des réseaux sociaux n'a fait qu'accentuer la défiance de la population vis-à-vis des pouvoirs publics. Comme l'a souligné le rapport, les sirènes d'alerte pour avertir la population sont totalement dépassées à l'heure où le Gouvernement peut informer directement nos concitoyens

en fonction de la nature de la crise- locale ou nationale -et des compétences de chacun. Ce retour d'expérience doit aussi nous permettre de mieux suivre l'activité des réseaux sociaux pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles.

des questions. Nous avons formulé dans notre rapport quarante propositions regroupées autour de six axes : la culture du risque ; la prévention ; la gestion de crise ; la coordination entre l'État et les collectivités locales ; l'indemnisation ; le principe de précaution. Je me réjouis également que le Gouvernement ait retenu un certain nombre de nos propositions dès le mois de février, et que certaines propositions complémentaires aient été émises

place un suivi épidémiologique, que nous appelons de nos voeux dans le rapport, sur une cohorte représentative des populations les plus impliquées dans la lutte contre l'incendie et ses conséquences.

; je parle sous le contrôle des élus de Seine-Maritime, notamment de ma collègue élue de Rouen. Ce qui préoccupe le plus la population aujourd'hui, ce sont les conséquences sanitaires de cette catastrophe à moyen et long terme.

Santé publique France, « les données sont très nombreuses, les formats restitués sont variés et il devient complexe d'avoir une analyse globale en vue d'en réaliser une synthèse ».

La séance est suspendue.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

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « des personnes en détresse, des enfants d'âge scolaire et des personnes ayant perdu durant les événements des derniers jours à Abidjan » : c'est dans ces termes que le Quai d'Orsay décrivait les Français évacués de Côte d'Ivoire lors des dramatiques événements politiques de 2004. Un coup d'État, un tremblement de terre, un tsunami, la prise de pouvoir par un groupe djihadiste, une pandémie sont des tragédies qui peuvent frapper les Français établis à l'étranger. Or aucun fonds d'urgence n'existe spécifiquement pour eux. C'est d'autant plus grave

La pandémie de covid-19 n'a fait que mettre en exergue à l'échelle mondiale une situation déjà connue depuis longtemps à l'échelon local, à savoir que nos compatriotes à l'étranger peuvent se retrouver du jour au lendemain dans un état de grand danger. C'est un révélateur. Le Gouvernement a réagi, mais en l'absence d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, il aura fallu aller chercher l'arbitrage de Bercy, ce qui nous a fait perdre un temps précieux. elle était adoptée, pérenniserait ce qui a été mis en oeuvre cette année, afin que dorénavant, lors d'une catastrophe naturelle ou sanitaire, ou lors d'un coup d'État, la réaction de la France soit immédiate pour venir en aide en urgence à nos compatriotes. Pourquoi un tel Pourquoi un tel fonds ? Quand un Français s'établit à l'étranger, il n'a souvent aucune garantie, aucun filet de sécurité. En cas de catastrophe, le retour en France se fait dans la précipitation, avec une valise, sans emploi, sans logement, et fréquemment avec des enfants. Une aide ponctuelle permet de rester sur place ou de retourner dans le pays après une évacuation temporaire vers la France, ce qui est la plupart du temps le souhait de nos compatriotes établis à l'étranger. à l'étranger. Je me souviens avec émotion des images, en novembre 2004, des 359 premiers Français évacués d'Abidjan, fuyant les violences en Côte d'Ivoire, arrivés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec une valise et des tongs au pied. Puis d'autres vols ont suivi pour évacuer plusieurs milliers de nos compatriotes, de manière temporaire ou définitive. Cette crise ivoirienne avait été précédée de nombreuses autres sur le continent africain. Ce sont notamment les guerres civiles des années 1990 en Afrique centrale, où les Français vivaient nombreux, qui avaient motivé les sénateurs des Français de l'étranger de l'époque pour tenter de créer un fonds de garantie. Les tremblements de Les tremblements de terre frappent aussi nos compatriotes à l'étranger. Je pense, par exemple, aux séismes survenus en 1999 à Izmit en Turquie, en 1988 en Arménie,

À l'avenir, il faudra également rester très vigilant pour les Français vivant dans les pays du G5 Sahel- Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad -, et qui sont confrontés au terrorisme islamiste. Le risque potentiel est immense pour nos communautés françaises, et un tel fonds d'urgence permettrait d'y faire face. La situation internationale ne prête pas à l'optimisme, car les conflits et les tensions Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, parle de « chaos ». Enfin, le dérèglement climatique et ses conséquences en termes de catastrophes naturelles font courir des risques nouveaux et de plus en plus nombreux.

Les consulats, par manque de moyens, doivent faire appel aux réseaux associatifs pour venir en aide à des familles en difficulté, car l'État ne le fait plus.

La crise de la covid-19 a été un révélateur de ce manque de moyens. Il a fallu intégrer un volet spécial pour les Français de l'étranger au plan global d'action visant à faire face à la crise sanitaire, mais on a perdu un temps précieux. Si le fonds d'urgence avait existé, les moyens auraient pu être mobilisés plus rapidement.

Comme me l'a rappelé Richard Yung, le groupe socialiste du Sénat avait lui aussi déposé une proposition de loi, sur l'initiative de notre ancienne collègue Monique Cerisier-ben Guiga. Joëlle Garriaud-Maylam en 2008 et encore à la fin du mois de mars cette année, ainsi qu'Olivier Cadic le 24 mars dernier, ont eux aussi déposé des propositions de loi.

Notre démarche s'inspire plutôt du Fonds de secours pour l'outre-mer ou du fonds d'extrême urgence pour les sinistrés des inondations, respectivement créés en 2012 et 2016.

d'inscrire notre texte à l'agenda du Sénat. Il démontre ainsi, une fois encore, sa compréhension des enjeux pour nos compatriotes établis hors de France, mais aussi pour la France. Je souhaite également rendre hommage au rapporteur de la commission des finances, Jérôme Bascher, dont la finesse d'analyse n'a d'égale que la capacité d'écoute. la création de ce fonds est dans l'intérêt de la France. Ce n'est absolument pas un cadeau fait aux expatriés. Contrairement aux idées reçues, les 3,4 millions de Français de l'étranger ne sont pas les abominables milliardaires déserteurs de la France et de sa fiscalité que l'on présente parfois.

pays. Nombre de ces Français paient des impôts et taxes- il existe d'ailleurs une direction des impôts des non-résidents -et leur participation au budget de l'État est tout à fait substantielle.

à une tragédie en restant dans le pays où ils sont établis, ou d'y retourner après un séjour provisoire en France, coûterait bien moins cher aux finances de l'État que leur réinstallation définitive en France, sans ressources, ni emploi, ni logement. Aucune politique de puissance n'existe sans le relais de compatriotes établis à l'étranger, qui oeuvrent pour le commerce extérieur, l'influence diplomatique ou le rayonnement culturel de leur pays. Nos compatriotes font partie intégrante de la Nation, même lorsqu'ils ne vivent plus en France. comme l'a dit le Général de Gaulle en 1967 : « Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut dissocier le sentiment et la politique. » La France doit démontrer le même attachement et le même amour à tous ses enfants, où qu'ils soient.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi de Ronan Le Gleut portant création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs.

ou encore les secours d'extrême urgence aux victimes d'accident, de sinistre ou de catastrophe de grande ampleur, mobilisés lors du passage de l'ouragan Irma ou des inondations dans l'Aude,

et au cas par cas et d'instaurer une doctrine d'attribution des aides d'urgence mobilisées lorsque les circonstances le nécessitent.

Ce fonds n'a, espérons-le, pas vocation à être souvent mobilisé. C'est la raison pour laquelle les conséquences budgétaires de sa création seraient, à la vérité, modestes

en France pour venir en aide aux Français victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves, telle la pandémie que nous connaissons, ou encore d'événements politiques majeurs, comme les guerres civiles ou les conflits. Ce texte est fondé sur le principe du secours, expression naturelle de la solidarité nationale, plutôt que sur le principe assurantiel, dont on sait que la mise en oeuvre peut être difficile ou tardive. Je tiens également à saluer le travail de la commission des finances, qui a

de traiter la plupart des pathologies de médecine générale, qu'elles soient aiguës ou chroniques, y compris en pédiatrie. Par ailleurs, 79 postes ont été équipés de lots comportant du matériel d'oxygénothérapie et des équipements de protection individuelle, afin de permettre la prise en charge de patients ayant besoin d'oxygène lorsque ce matériel est peu ou pas disponible. Au total, 11 générateurs et 128 extracteurs d'oxygène avec les consommables nécessaires ont été envoyés. Cela mérite d'être signalé. Une cinquantaine de postes sont à ce jour dotés de tous ces matériels. En outre, un mécanisme d'évacuation sanitaire a été mis en place, avec des avions dédiés,

il permet une véritable solidarité nationale, grâce à un certain nombre d'allocations, une aide au rapatriement, un soutien aux associations françaises locales de bienfaisance à l'étranger. Chaque année, près de 17 millions d'euros sont consacrés à nos compatriotes les plus en difficulté, à travers une gamme d'allocations ciblées. Je pense à

Leur éloignement géographique de la France peut les priver d'un certain nombre de dispositifs de protection devenus indispensables et mis en oeuvre dans notre propre pays. L'État, comme l'a dit Ronan Le Gleut, leur doit pourtant la protection, comme à tout citoyen français,

Le Gouvernement a déployé des efforts exceptionnels pour les Français qui étaient à l'étranger au début de la crise, mais les rapatriements ont visé principalement les Français de passage, alors que les résidents installés sont, eux, restés sur place.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la sagesse populaire nous dit que c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis. Je crois que c'est également à cette aune que les Français jugent l'action publique : c'est dans le besoin que l'on reconnaît le véritable rôle de l'État. De ce point de vue, la crise sanitaire a fait l'effet d'un révélateur : les Français ont ainsi reconnu, si besoin en était, l'importance d'un État fort et robuste. De fait, l'État a tenu bon, malgré des conditions économiques et sanitaires extrêmes. Cela vaut pour tous les Français, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières. Aider nos concitoyens à l'étranger s'avère aussi nécessaire que délicat, en temps de crise plus encore que de coutume. La puissance publique doit constituer pour eux un appui et une garantie sans faille, d'autant plus lorsque les relations internationales se crispent face aux tensions sanitaires. Nombre de nos concitoyens établis hors de France ont pu compter sur un État réactif et agile, qui a su s'adapter à des contextes étrangers très variés. Je crois que ce sentiment est très largement partagé, et je tiens à le signaler. Le crédit en revient en partie au Gouvernement, mais aussi, pour une grande part, à notre réseau diplomatique, qui a de nouveau fait la preuve de son efficacité et de ses compétences. Lorsqu'une crise survient, qu'elle soit sanitaire, sociale ou politique, on est en droit d'attendre que le Gouvernement prenne les mesures adaptées, car il échoit à l'exécutif de répondre à l'urgence d'une situation par l'action. Mais cette intervention ne se déploie jamais que dans le cadre voté par le Parlement. C'est pourquoi je salue l'initiative de Ronan Le Gleut, qui vise à construire le cadre d'une intervention adaptée à des situations d'urgence par la création d'un fonds destiné à cette finalité. Il s'agit d'une bonne solution pour préparer aujourd'hui les interventions de demain, qui devront nécessairement pouvoir avoir lieu sans attendre. À l'heure où nous examinons ce texte, la menace sanitaire n'a pas disparu, mais nous aurions tort d'aborder cette proposition de loi comme un texte de circonstance. D'ailleurs, la création de ce fonds est une idée qui a fait son chemin. La crise aura donc tout au plus joué le rôle de catalyseur dans le processus législatif.

mais ces dispositifs ne sont bien évidemment pas calibrés pour des situations exceptionnelles comme celle que nous avons connue. Aussi, je crois utile que nous instaurions un mécanisme général destiné, par nature, à subvenir à des besoins particuliers. Je n'y vois aucune contradiction : c'est le principe même de tout mécanisme assurantiel. Le chiffre annoncé de 30 millions d'euros d'abondement annuel semble raisonnable, compte tenu des montants mobilisés lors des dernières interventions d'urgence auprès de nos concitoyens à l'étranger. Des ressources complémentaires pourraient également être puisées dans la réserve de précaution en cas de crise majeure, ce qui permettra d'articuler prévoyance et souplesse. Je vous proposerai une autre source de financement alternative, avec l'augmentation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Nous aurions pu également envisager la majoration de 10 % du tarif des passeports. J'espère que le débat nous permettra d'identifier ensemble le modèle de financement le plus adapté. En tout état de cause, cette proposition de loi contribue à rendre plus lisibles les efforts réalisés par la Nation en faveur de nos concitoyens établis hors de France. il semble pertinent de distinguer les aides exceptionnelles d'urgence versées en cas de crise majeure des aides de droit commun. C'est l'une des ambitions de ce fonds,

C'est pourquoi les amendements qui ont été adoptés sur le texte initial par la commission des finances vont dans le bon sens. Ils visaient non pas à restreindre le champ d'application du fonds, mais bien à préciser les situations dans lesquelles celui-ci pourrait être mobilisé. Mon groupe s'y montre également favorable. De la même manière, nous considérons qu'il est plus pertinent de ne pas caractériser de façon superfétatoire les aides qui pourraient être versées par le biais du fonds. Encore une fois, il ne s'agit en rien de restreindre la portée de l'action de celui-ci : l'objectif est bien d'en sécuriser les interventions. C'est, je crois, soutenir son ambition initiale. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants apporte son soutien à cette proposition de loi. Améliorer l'efficacité de l'action publique, clarifier l'emploi des ressources publiques, renforcer le rôle de l'État en France comme à l'étranger, agir en prévention des catastrophes à venir, en prenant notamment les devants face au dérèglement climatique : nous

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je félicite chaleureusement Ronan Le Gleut pour son initiative, qui nous amène à débattre de la création d'un fonds d'urgence pour les Français établis à l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques graves. Depuis des décennies, l'Assemblée des Français de l'étranger l'appelle de ses voeux.

tous ces efforts se sont révélés vains. Les gouvernements successifs, quelle que soit leur appartenance politique, ont toujours opposé des motifs budgétaires pour justifier l'impossibilité de créer un un fonds public d'indemnisation faisant appel à la solidarité nationale. Je veux donc saluer l'action de notre rapporteur pour trouver une solution, afin de rendre possible ce que tant attendent. Ne pas disposer d'un fonds pour aider nos compatriotes établis à l'étranger victimes de catastrophes naturelles nous condamne à l'impuissance lorsqu'un drame survient. Tannya Bricard, conseillère consulaire en Équateur, l'a constaté lorsqu'elle recherchait du soutien pour nos compatriotes affectés par le tremblement de terre de 2016, qui a fait plus de 1 000 victimes dans son pays d'adoption qui a notamment ravagé la ville de Manta, dans laquelle elle vit. Je me suis rendu à Manta l'an dernier. J'y ai rencontré ces Français, qui m'ont dit qu'ils avaient été oubliés par notre Tous nos compatriotes déploraient que la France ne leur ait offert aucune assistance pour faciliter le redémarrage de leurs activités. Chacun témoignait que seule l'aide de leur famille et de leurs amis leur avait permis de se relancer le cas échéant. Au moment de soutenir le texte présenté ce jour, je pense à Tannya et à nos compatriotes de Manta. Je pense à Martine, productrice de crevettes. Ses bassins et diverses infrastructures s'étalaient sur 100 hectares. Tout a été dévasté. Je pense à Thierry, capitaine de pêche thonier, qui m'a accueilli dans le restaurant de sa femme en me faisant observer que le restaurant péruvien situé à proximité avait reçu, lui, une aide du Pérou pour redémarrer. à Christian, qui avait ouvert un bar-restaurant en Équateur et qui, après le séisme, ne savait plus où habiter. Je pense à Émilie, qui avait démarré une usine de purification d'eau pour pallier un problème sanitaire. Je pense jeune boulanger pâtissier qui s'était lancé à Manta deux ans plus tôt. Pendant une année, il n'a pas pu travailler, passant son temps à remplir de la paperasse pour décrocher un prêt bancaire ou une aide d'un organisme qui avait recueilli, lui, des fonds de l'Agence On imagine le triste sentiment qu'ils éprouvaient, celui de ne pas avoir été pris en compte par leur pays et de ne devoir alors compter que sur eux-mêmes et sur leurs proches. En ce moment, je pense également à Jean-Louis Mainguy, conseiller consulaire Liban-Syrie, qui, en décembre 2019, alertait sur l'impérieuse nécessité de venir en aide aux Français du Liban. La crise exceptionnelle traversée par ce pays a plongé 45 % de la population au-dessous du seuil de pauvreté, dont nombre de Français. Le 17 mars Le 17 mars dernier, Jean-Louis Mainguy, également vice-président de l'UFE Monde et administrateur de la Caisse des Français de l'étranger, a d'ailleurs décidé d'écrire au Président de la République pour lui demander justement d'instaurer un fonds permanent de solidarité et d'entraide. de février dernier, tandis que j'étais en Égypte, la conseillère consulaire Régine Prato, présidente de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens à

pressé par la pandémie naissante, j'avais intégré la création d'un tel fonds à ma proposition de loi relative à la solidarité en faveur des Français établis à l'étranger en période de crise, déposée le 24 mars dernier. dernier. Il n'y a aucune raison que la solidarité nationale s'arrête à nos frontières. À l'époque, l'urgence était de faire face à la crise sanitaire mondiale. J'avais donc proposé que les Français expatriés bénéficient eux aussi du fonds de solidarité créé par la loi d'urgence du 23 mars 2020 tout spécialement pour faire face à l'épidémie de covid-19. C'était l'objet de l'article 1 de ma proposition de loi, qui, je dois le dire, a été pleinement satisfait. En effet, le 30 avril dernier, par votre voix, monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement annonçait un plan de soutien de 220 millions d'euros en faveur de nos compatriotes résidant à l'étranger.

Mais, si l'article 1 de ma proposition de loi concernait le court terme, l'article 2 visait à créer un fonds d'urgence et de solidarité pour secourir nos compatriotes victimes de circonstances graves. C'est pourquoi je me retrouve pleinement dans l'initiative de Ronan Le Gleut et de ses cosignataires. Il est important que nous soyons rassemblés au-delà des clivages pour être efficaces et faire aboutir ce texte. Je remercie tous les parlementaires qui se sont associés à ma démarche, en particulier les sénateurs représentant les Français établis hors de France Robert del Picchia, Damien Regnard et Richard Yung.

Cela va sans dire ! Pour moi, la question est : quand ? Avant leur attribution ? Après celle-ci, comme nous l'observons actuellement dans la procédure d'attribution des 50 millions d'aide sociale d'urgence ? j'ai eu l'opportunité de le dire par le passé, le Gouvernement sera aussi jugé sur sa capacité à répondre à l'urgence sociale que vivent nos compatriotes à l'étranger. Il cherche à se donner les moyens d'y répondre vite, et c'est heureux. Reste à garantir que ces moyens seront tous orientés vers la finalité recherchée. Il est donc impératif que les postes diplomatiques s'appuient instamment sur les conseillers consulaires pour construire les plans de soutien et organiser l'attribution des aides directes ou indirectes. Il en irait de même dans l'organisation de l'attribution de l'aide émanant du fonds proposé.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les Français de l'étranger font pleinement partie de la communauté nationale, comme le rappelait Jérôme Bascher. Même loin des yeux, ils ne sont jamais loin du coeur. du coeur. Tout comme ceux qui résident sur le territoire national, ils ont été durement touchés par la crise sanitaire que nous sommes encore en train de vivre. Cette situation a révélé un manque, dans nos outils de politique publique, pour faire face à une situation exceptionnelle. Bien évidemment, je le dis sans remettre en cause le travail admirable effectué par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour venir en aide à nos à nos compatriotes. Pour pallier ce manque d'un outil de politique publique, qui est relevé depuis longtemps, le texte dont nous discutons aujourd'hui, sur l'initiative de Ronan Le Gleut, prévoit l'institution d'un mécanisme d'urgence pour aider des Français qui peuvent, n'importe où dans le monde, être confrontés à des catastrophes naturelles ou à une menace sanitaire. Il est vrai qu'aucun fonds spécifique n'existe à à cet effet. Nous devrons voter des crédits dans le cadre du projet de loi de finances rectificative dans quelques jours. Si elle est retenue, la présente initiative montrerait la volonté de la France de secourir tous ses ressortissants, où qu'ils se trouvent. Si sa mise en oeuvre reste encore assez floue, disons-le clairement, nous partageons cette volonté. Nos collègues représentant les Français établis hors de France nous alertent depuis longtemps déjà sur le manque de moyens alloués aux consulats et ambassades pour venir en aide à nos concitoyens à l'étranger. Ils ne manquent pas d'exemples pour montrer la nécessité d'accroître nos moyens d'intervention.

chers collègues, à l'approche d'élections consulaires et sénatoriales finalement reportées de quelques mois ... La période que nous traversons actuellement, avec la crise sanitaire, qui, dans la plus grande partie du monde, est bien loin d'être terminée, montre à quel point la préoccupation qui nous anime est légitime. La pandémie a obligé l'État à dégager des moyens exceptionnels, que nous allons être amenés à inscrire dans la loi de finances : 50 millions d'euros pour aider les familles ayant connu une baisse importante de leurs revenus et ne pouvant plus payer les frais de scolarité 50 millions d'euros pour permettre aux ambassades, consulats et associations de venir en aide aux Français de l'étranger les plus démunis, qui ne reçoivent pas d'aide de la part de leur pays de résidence ; 20 millions d'euros pour suivre et conseiller au niveau médical les expatriés français les plus vulnérables

Cette proposition de loi a, par conséquent, un défaut : nous ne connaissons pas, à ce stade, le coût qu'elle représenterait pour les finances publiques. Le mois nous avions déjà soulevé cette absence d'évaluation chiffrée des mesures contenues dans la proposition de loi du groupe Les Républicains. Cela dit, est-il possible de faire différemment ? Le vote d'un budget relève de toute façon d'une loi de finances Nous approuvons la création de l'outil, celui d'un fonds d'urgence, et non d'un fonds d'indemnisation. Cette dimension de secours, qui ne relève pas d'une logique assurantielle, a été clarifiée par la suppression, en commission des finances, du deuxième alinéa de l'article 1. Je pense que c'est une bonne chose. Le devenir de cette proposition de loi reste bien sûr encore assez aléatoire. Toutefois, elle a d'ores et déjà un mérite : nous inviter et inviter le Gouvernement à pérenniser des réponses qui doivent être trouvées en urgence cette année face à la crise sanitaire. C'est pourquoi, sous réserve des conclusions de notre débat, les membres du groupe socialiste et républicain approuveront très probablement ce texte. La parole

mais que la crise du covid-19 a remise en lumière. Il s'agit de répondre, par l'institution d'un instrument pérenne, aux situations d'urgence qui peuvent affecter nos concitoyens établis hors de France. Certains de nos collègues ont déjà, par le passé, pris des initiatives pour créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. On doit bien comprendre que l'action de l'État peut se diluer avec la distance. Bien que les expatriés disposent de droits et d'institutions à leur service, l'isolement et l'éloignement du pays d'origine ne facilitent pas l'assistance en cas de crise. Si la situation de confinement a été une épreuve pour nous tous, elle a parfois été plus violente dans certains pays, en fonction des règles adoptées par ceux-ci. C'est pourquoi plusieurs problèmes spécifiques se sont posés pour nos concitoyens éloignés. Je pense, en particulier, à l'incidence de la fermeture des frontières et d'espaces aériens, qui a coupé les relations familiales. Je songe aussi à la dégradation de la situation économique, qui a plongé des foyers français dans la détresse. La crise sanitaire a également mis les établissements d'enseignement français à l'étranger en grande difficulté, des parents ne pouvant plus payer les frais de scolarité. Enfin, je n'oublie pas la question des frais médicaux qu'a pu soulever l'épidémie de façon inattendue. Monsieur le secrétaire d'État, nous savons bien que l'État n'est pas resté sourd à ces difficultés. On peut, en particulier, saluer l'action des postes consulaires, qui se sont démenés pour faire face, avec des moyens limités. Dans l'urgence, le Gouvernement a mis sur pied un plan de soutien de 50 millions d'euros, engagés au sein du programme budgétaire consacré aux Français à l'étranger et aux affaires consulaires. Par ailleurs, la revalorisation de l'enveloppe des aides à la scolarité a permis d'assurer la continuité pédagogique pour des milliers d'élèves. À la lumière de cet événement et des retours de terrain qu'ont pu avoir nos collègues élus de l'étranger, il apparaît clairement nécessaire de créer un fonds suffisamment alimenté et réactif pour éviter un secours désordonné ou trop tardif. Contrairement aux idées reçues, nos concitoyens vivant hors de nos frontières ne sont pas que de riches expatriés ou des exilés fiscaux, comme l'ont d'ailleurs comme l'ont d'ailleurs rappelé les orateurs précédents. Parmi ces 2,5 millions de Français, il y a des gens modestes et des retraités aux petites pensions, dont la situation peut vite se dégrader. M. le rapporteur a rappelé le système actuel d'aides directes ou indirectes pour les personnes socialement ou économiquement fragilisées. Existent, en particulier, des aides ponctuelles. Ces dernières, de l'allocation à durée déterminée, de l'aide sociale à l'enfance ou des secours occasionnels, permettent d'apporter des réponses à petite échelle, mais s'avèrent insuffisantes en cas de crise ou de catastrophe de grande ampleur. On l'a constaté notamment à l'occasion de la crise du covid-19. Aussi, mon groupe est favorable à la création d'un fonds d'urgence qui serait complémentaire des dispositifs actuels et surtout mobilisable en cas de menaces sanitaires graves, de catastrophes naturelles, de guerres civiles ou étrangères et de révolutions. Cet instrument s'inspire du fonds pour l'outre-mer. C'est une bonne chose. La commission des finances a apporté quelques correctifs à la marge, en particulier la suppression de la subrogation pour l'État dans les droits de tout bénéficiaire. J'approuve cette démarche. En effet, toute action récursoire à l'encontre d'un État ou d'une personne privée de droit étranger serait vaine et, en tout cas, très compliquée, à moins d'un accord bilatéral. S'agissant de la procédure d'attribution, l'inscription, dans le marbre de la loi, de la condition de ressources est nécessaire pour mieux conforter le caractère solidaire du fonds. À ce stade demeure toutefois une inconnue. Quel type de financement apporter et à quel niveau ? J'espère que le présent débat permettra de lever quelques-unes des interrogations sur la mécanique financière de ce fonds d'urgence. En attendant, mes chers collègues, le RDSE approuvera la proposition de loi,

des Français établis hors de France, qui, en particulier en ce moment, sont nombreux à subir de plein fouet la pandémie et ses conséquences. Je veux aussi remercier le Gouvernement des mesures de soutien qu'il a prises pour faire face à cette pandémie, que le troisième projet de loi de finances rectificative va nous permettre d'adopter. L'abondement de l'enveloppe des aides sociales consulaires et l'augmentation des crédits vont nous permettre de répondre aux besoins. Le redéploiement des crédits en faveur des organismes locaux d'entraide et de solidarité

Deux mois jour pour jour après la présentation du dispositif de soutien, nos collègues de la majorité sénatoriale proposent que les mesures de soutien aujourd'hui financées par un collectif budgétaire ou un redéploiement de crédits soient, à l'avenir, mises en oeuvre la mobilisation d'un fonds d'urgence, alimenté par le budget de l'État et qui, contrairement aux autres fonds de même nature, disposerait d'un fondement législatif.

le plus souvent sous l'angle de l'indemnisation des dommages subis à l'étranger. L'objectif était alors de tirer les conséquences d'événements tragiques, comme la crise ivoirienne ou le conflit israélo-libanais. Je rappelle ainsi que le rapatriement de 8 000 Français de Beyrouth Beyrouth avait été une grande opération. Les mécanismes d'indemnisation proposés reposaient soit sur le principe de la solidarité nationale, soit sur celui de l'assurance. Pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, j'ai souvenir d'avoir entendu Nicolas Sarkozy proposer la création d'un « fonds d'assurance indemnisation des Français spoliés son appellation -lors de conflits ou de catastrophes naturelles, mais cette promesse n'a pas été suivie d'effet. J'avais alors déposé une proposition de loi visant à améliorer le régime d'indemnisation des dommages subis à l'étranger. Le dispositif que j'avais en tête était mixte. J'avais en effet proposé de faire appel à la solidarité nationale pour l'indemnisation des dommages corporels et de conjuguer la solidarité nationale et l'assurance pour l'indemnisation des dommages matériels. Il s'agissait concrètement de rajouter 0,01 % aux primes d'assurance qui servent à financer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

La crise que nous traversons montre la nécessité de subvenir rapidement aux besoins de première nécessité. C'est pourquoi je trouve judicieuse l'idée d'emprunter la voie du secours que propose Ronan Le Gleut et de créer un vecteur pérenne de l'aide d'urgence. Ce mécanisme relève du bon sens. Il permettra de réduire les délais dans lesquels les crédits d'urgence sont mobilisés et complétera le dispositif de gestion de crise du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont nous avons pu constater la grande efficacité durant la dernière crise. Par ailleurs, subordonner l'accès au fonds à une inscription au registre

serait de nature à inciter nos ressortissants à s'enregistrer auprès de leur consulat, à commencer par ceux qui se trouvent dans des pays difficiles. Pour que ce fonds d'urgence puisse rapidement être activé, il conviendra de lui allouer une dotation en loi de finances. C'est ce qu'a excellemment prévu et développé le rapporteur, et je fais mienne sa proposition d'une dotation d'au moins 30 millions d'euros, soit 20 millions d'euros de plus que la dotation du fonds de secours pour l'outre-mer. d'appeler votre attention sur la nécessité de placer cette réflexion dans le cadre européen. Selon moi, il serait utile d'étudier la possibilité d'élargir le champ d'application du Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui a été créé pour faire face à ces grandes catastrophes.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est bien la maison des Français de l'étranger. Nous en avons eu un très bel exemple le 19 mai dernier, lors de l'adoption de la proposition de loi de Bruno Retailleau, dont j'étais rapporteur, qui a trait à la plupart des sujets que nous défendons tous sur ces travées de façon transpartisane depuis un bon nombre d'années. fallait cependant aller plus loin pour que les Français résidant hors de France soient rétablis dans leur appartenance à leur patrie, pour qu'ils soient des Français à part entière et plus jamais des citoyens de seconde zone.

représentant les Français de l'étranger ont toujours répondu présent, quel que soit leur groupe politique, pour soutenir nos compatriotes expatriés lors des nombreuses catastrophes naturelles et crises qu'ils ont dû affronter. Ils l'ont toujours fait en lien étroit avec les acteurs de terrain que sont les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, les délégués consulaires. Merci à Ronan Le Gleut d'avoir encore une fois pensé à eux. Dans le monde très agité où nous vivons, où le terrorisme n'a pas désarmé, où, parfois, la nature s'emballe, où des conflits surgissent, nous essayons depuis longtemps de trouver une solution qui puisse être immédiatement activée sans avoir à attendre des décisions souvent trop longues à se mettre en place. Cette proposition de loi ouvre un champ très large sur les événements concernés : crise sanitaire ou économique, catastrophes naturelles, guerre civile ou étrangère, toutes les situations sont visées. À ce jour, il existe plusieurs fonds d'urgence spécifique en France et en outre-mer. Jusqu'à présent, les Français établis hors de France ont seulement droit au fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui s'applique indifféremment à tous les Français. Les Français résidant hors de France ne peuvent prétendre à aucun autre soutien, contrairement à leurs compatriotes de métropole et d'outre-mer. Il est donc urgent de créer un fonds pour eux qui, partout dans le monde, portent les belles couleurs de notre drapeau, qui sont fiers d'être Français, qui ont fait la preuve qu'ils étaient courageux, qui ne bénéficient pas des aides sociales- chômage, retraite, sécurité sociale, école gratuite ... -et tant d'autres avantages réservés aux Français qui vivent dans l'Hexagone ou outre-mer. Ils ne souhaitent qu'une chose, ne jamais avoir à tendre la main, mais il y a des circonstances où la nature, la politique, les virus vous font trébucher et, sans une main qui se tend, on ne peut pas se relever et on s'effondre. Ils n'auront besoin de notre solidarité que pour les aider à passer une vilaine vague, quelques mois seulement, et ils repartiront et seront de nouveau ces gens courageux dont nous sommes si fiers. Ce fonds est un fonds de secours qui n'a vocation à être utilisé que dans des circonstances très particulières. Cette proposition de loi pose des principes de base et renvoie les mesures d'application au Gouvernement, lequel, sur le fondement des informations des postes diplomatiques et consulaires, dont le dévouement est unanimement reconnu, et des informations des élus des Français de l'étranger, est le plus à même de trouver les solutions les plus adaptées. Je me réjouis que le rapporteur, Jérôme Bascher, ait proposé un amendement reprenant l'objet de celui que j'avais déposé sur les conseils consulaires et l'ait fait adopter par la commission des finances. à prévoir la consultation des conseils consulaires pour l'octroi des aides dans le cadre du fonds d'urgence. Mes chers collègues, pour la deuxième fois en quelques semaines- ce qui n'était pas arrivé depuis si longtemps -, tous ensemble, redisons à nos compatriotes qui vivent loin de nous que nous ne les abandonnerons pas, où qu'ils soient, quoi qu'il leur arrive. Nous continuerons à marcher côte à côte. Ceux qui vivent à l'étranger aiment la France, ils y ont leurs racines, leur famille, leurs amis. Pour ceux qui vivent en France, dans l'Hexagone ou en outre-mer, les Français résidant à l'étranger sont leurs dignes représentants, ceux qui portent notre voix aux quatre coins du monde. Ils font connaître notre langue, notre culture, nos produits. Tous ensemble, nous sommes la France dans sa plus belle diversité, avec nos accents, nos coutumes, nos paysages tous différents, mais rassemblés et unis sous le même drapeau.

Notre lointain prédécesseur, qui siégeait dans cet hémicycle il y a un siècle et demi, l'immense poète Victor Hugo, me pardonnerait, je l'espère, le détournement de son magnifique poème. Il comprendrait peut-être, lui qui vécut l'exil, mon désir de rendre hommage à tous ces femmes et hommes qui vivent loin de leur mère patrie, tout en y restant profondément attachés. Il nous faut casser l'image totalement fausse du Français de l'étranger exilé fiscal, image complaisamment entretenue dans les bureaux feutrés de certains ministères- pas le vôtre, monsieur le secrétaire -ou véhiculée par des journaux à sensation qui nous exhibent les photos de la luxueuse villa de telle star du show-business ou du football, partie vivre sous des cieux fiscalement plus cléments que le nôtre. Sur les 3,5 millions de Français établis hors de France, combien sont-ils, ces exilés fiscaux, sinon quelques centaines, quelques milliers tout au plus ? Les autres, tous les autres, sont aussi divers que les Français de France ! Fort de toutes ces années à voyager et à les rencontrer, je peux en témoigner. De l'enseignant au restaurateur, du jeune qui a raté ses études et qui est parti comme serveur dans un pub au cadre d'entreprise, du retraité à l'avocat, du boulanger au médecin, en passant par le responsable d'ONG, ils sont la France et font rayonner notre Comme les Français de France, ils peuvent subir de plein fouet les tragédies de la vie, mais, contrairement aux Français de France, ils n'ont aucune garantie et peuvent se retrouver du jour au lendemain dans la détresse la plus absolue, sans chômage, sans aide, sans rien De constat en constat, d'intervention en intervention, les urgences affluent. Tout a été dit sur un sujet aussi brûlant que celui de l'aide d'urgence à apporter à nos compatriotes en cas de crise. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la volonté de trouver un mécanisme permanent de réponse aux situations d'urgence comme celle que nous vivons en ce moment. La proposition de loi que, sous l'impulsion de Ronan Le Gleut, nous avons déposée le 10 février dernier se situe dans la lignée de précédentes initiatives. Je me souviens avec émotion que nos anciens collègues Paulette Brisepierre, Charles de Cuttoli, Jacques Habert et tant d'autres avaient déjà déposé en 1990 et en 1998 une proposition de loi portant création d'un fonds de solidarité. Joëlle Garriaud-Maylam a également déposé une proposition de loi portant création d'un fonds de solidarité en 2008,

relative à la solidarité en faveur des Français établis à l'étranger, considérant l'état d'urgence sanitaire mondial. La mobilisation est donc générale. Il faut la saluer- aucune rivalité ni ego. Il revient cependant à notre collègue Ronan Le Gleut d'avoir compris le premier cette année le désastre qui se préparait à l'échelle mondiale, avec ses conséquences pour les Français de l'étranger, et combien il devenait nécessaire de mettre en place un mécanisme d'urgence pérenne. Cette proposition de loi a le mérite d'être la première à s'inspirer de ce qui existe déjà en France, à savoir le fonds d'urgence pour l'outre-mer ou encore le fonds d'extrême urgence pour les inondations, avec un mécanisme souple pouvant être activé sans délai. Il s'agit ici de mettre en place, dans les cas de catastrophe naturelle, de menace sanitaire grave ou d'événement politique majeur, ce même type de dispositions pour nos compatriotes de l'étranger, qui, je vous le rappelle, sont par ailleurs contribuables et participent eux aussi, par diverses contributions, à la solidarité nationale. Un formidable travail de remodelage a été réalisé par notre rapporteur Jérôme Bascher, dont je salue l'intérêt et la compréhension envers les sujets touchant les Français de l'étranger. Je tiens aussi à remercier chaleureusement le président Bruno Retailleau, grâce auquel nous examinons aujourd'hui, dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe Les Cette proposition de loi est désormais une évidence et l'actualité justifie amplement son adoption. Un plan d'urgence a été mis en place pour nos compatriotes de l'étranger, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État. Les fonds débloqués ont tardé à venir, car le mécanisme n'existait pas. Si le fonds avait déjà existé, je pense que Pensons à l'avenir et aux prochaines crises sanitaires, naturelles ou politiques, qui, hélas, ne manqueront pas de survenir. La proposition de loi de Bruno Retailleau qui a été votée voilà quelques jours a consacré un certain nombre de mesures dont nous souhaitions depuis plusieurs années

quoi qu'il en coûte ». Au contraire, ce fonds est lié au texte que nous venons d'adopter visant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure. Si tant de mesures sont prises en France, aujourd'hui, pour répondre aux situations imprévues et aux catastrophes, pourquoi ne pas les étendre de manière durable à nos compatriotes de l'étranger, qui, un jour, ont été, sont ou seront victimes d'événements aussi violents qu'imprévus

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les Français établis hors de France, dont nous parlons beaucoup au Sénat depuis quelques mois, alors que notre rendez-vous annuel est généralement au mois de novembre lors de la discussion budgétaire, représentent une population aussi diverse dans ses origines et sa composition que celle de la France. Chaque histoire est différente, les motifs de l'expatriation sont intimes à chacun d'entre eux. Plus que d'autres, ces Français établis hors de France ne peuvent se résumer en une catégorie qui rassurerait et en faciliterait la compréhension. Avec eux, il est difficile de cocher des cases, parce qu'ils n'y entrent pas facilement. Chaque parcours, chaque histoire est irréductible à l'autre. Par-delà la caricature facile et injuste, ces Français de l'étranger nous disent cependant tous quelque chose de nous-mêmes et de la France. Vus d'ailleurs, notre identité, notre influence, nos qualités et nos défauts apparaissent ou se relativisent, se grandissent et se fondent. Partis trop longtemps ou nés à l'étranger, mais revendiquant toujours leur identité française, ils sont confrontés au choc culturel ressenti à chaque changement de lieu parce qu'ils sont devenus « l'autre » et sont perçus comme tels par leurs compatriotes. Mal connus et mal aimés, la stigmatisation dont ils sont les cibles relève d'une méconnaissance de cette communauté hétérogène et repose sur les clichés d'une autre époque d'une population oisive et fortunée. Il est par ailleurs intéressant de noter que nombre de Français vivant à l'étranger refusent le terme d'expatriés, ... C'est vrai ! ... qui ne correspond pas à leur statut, en tout cas à ce qu'ils perçoivent être la définition de ce terme auquel sont associés des privilèges. Cet état de fait sémantique est révélateur de son évolution, qui a introduit une dimension humaine fondamentale. Elle nie également pour ces derniers le mérite d'une démarche qui, au contraire, atteste que la France s'inscrit dans le monde on semble avoir oublié que l'envie de se déplacer a toujours existé pour aboutir à la découverte de nouveaux mondes et jusqu'à celle de l'espace. Son accélération est une réalité dont les Français font aujourd'hui partie : la mondialisation ne s'est pas arrêtée aux frontières de la France et la crise que nous traversons nous le rappelle quotidiennement. Plus de 3,5 millions de Français vivent aujourd'hui à l'étranger, montrant ainsi que nous sommes une nation ouverte, reconnue et appréciée. En outre, où qu'ils soient sur la planète, les Français se sentent toujours des Français à part entière. Représentant 5 % de la population française, il est légitime qu'ils soient représentés au Parlement et localement. La loi du 7 juin 1982 introduisant le suffrage universel dans la représentation de nos compatriotes expatriés avait été défendue avec passion et résolution par Claude Cheysson. ans plus tard, animée des mêmes sentiments, j'avais repris cette réforme modifiant la représentation politique des Français de l'étranger dans le sens d'une plus grande équité, d'une plus grande proximité et d'une plus grande vitalité citoyenne. Tel a été mon objectif en 2013. Grâce à l'élection de 443 conseillers consulaires au mois de mai 2014, les Français de l'étranger disposent désormais de l'écoute et de la reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre. La crise actuelle montre combien leurs élus locaux sont précieux dans l'information et le soutien qu'ils apportent aux plus vulnérables. Ils connaissent parfaitement la situation des familles. S'il est adopté, l'amendement déposé par mon groupe leur accordera la place qui doit leur revenir dans un dispositif d'octroi d'une nouvelle aide financière qui complétera les aides accordées par l'État. Celles-ci sont actuellement allouées par les conseillers consulaires sur la base de critères bien définis et sont restreintes à l'éducation et au social. Les crises politiques, climatiques ou sanitaires sont nombreuses ; elles précarisent bon nombre de nos compatriotes, notamment nos entrepreneurs implantés de longue date dans leur pays d'accueil, présents dans le monde entier.

Je salue donc le texte qui nous est soumis aujourd'hui par notre collègue Ronan Le Gleut et son groupe et qui vise à venir en aide à nos compatriotes établis hors de France. Si le concept n'est pas nouveau, cela a été rappelé, il est cependant bienvenu et tombe à point.

La France a encore des difficultés à valoriser son implantation planétaire hors du commun. Elle doit chercher toujours plus à accompagner ses compatriotes et à faire preuve de solidarité. Ce fonds montrera vite sa grande utilité, notamment pour les recrutés locaux et les contractuels, quel que soit leur domaine d'activité dans nos ambassades, établissements scolaires, alliances françaises, instituts français, ou nos entrepreneurs et artisans, pour leur permettre de traverser les crises qui frappent leur pays de résidence sans être forcés à le quitter.

pour louer nos compatriotes de l'étranger. Bien évidemment, je partage leurs propos et tiens à remercier notre ministre des affaires étrangères de son action inlassable en faveur des Français de l'étranger pendant cette crise. Je regrette cependant que ma proposition d'aide aux tout petits entrepreneurs français de l'étranger dans le cadre du fonds de solidarité aux entreprises ait été refusée

Ainsi, l'exposé des motifs indique que, depuis plus de deux décennies, des sénateurs des Français de l'étranger ont rédigé des propositions de loi tendant à créer des fonds d'indemnisation pour les Français résidants à l'étranger dans une logique assurantielle.

en 2016, je tiens à le préciser parce que cela a été oublié dans les interventions, après la crise en Équateur mentionnée par Olivier Cadic et pour laquelle j'avais mobilisé ma réserve parlementaire,

et taxes sur les passeports. C'est celle-ci qui, de toute évidence, a inspiré Ronan Le Gleut, puisque, en 2017, alors qu'il était candidat dissident avec le soutien de l'UDI contre moi, il intégrait cette proposition de fonds de solidarité dans ses promesses électorales.

Comme l'a dit avec humour une collègue de la commission des finances lors de l'examen du rapport : ces deux textes, ce sont un peu les mêmes raviolis, c'est juste l'étiquette de la boîte qui change !

Lepage, sur l'article. « Vous êtes les ambassadeurs de la France. » C'est en ces termes que les Présidents de la République, tous bords confondus, les ministres des affaires étrangères et autres ministres saluent la communauté française lors de leurs déplacements à l'étranger. Aucun d'entre eux ne manque d'évoquer devant les entrepreneurs français, les représentants d'association et les membres de la communauté française présents l'importance des Français établis hors de France pour le rayonnement de notre pays. Cependant, si une catastrophe naturelle survient- séisme, éruption volcanique, tsunami si une crise politique grave surgit, amenant son lot d'exactions et de pillages, si une crise sanitaire se déploie, rien n'est prévu pour les aider, eux qui ont perdu leurs biens, leur outil de travail, et qui se retrouvent démunis. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, devenu Assemblée des Français de l'étranger en 2004, avait en son temps, comme vous l'avez déjà entendu, travaillé sur le sujet pour proposer la mise en place d'un fonds de solidarité afin d'aider nos ressortissants en cas de catastrophe. Deux voies étaient possibles : la piste assurantielle ou la création d'un fonds d'urgence garanti par l'État. La solution l'assurance s'est vite révélée trop onéreuse pour nos compatriotes et les gouvernements successifs n'ont pas voulu s'engager sur la voie d'un fonds garanti par l'État. La proposition de loi de Ronan Le Gleut va donc dans le bon sens et je l'en remercie. Certes, le Gouvernement a déployé des efforts importants pour faire face aux difficultés liées à la crise du covid-19 pour les Français de l'étranger, mesures que nous devrons voter prochainement, mais la création d'un fonds d'urgence permettra de réagir rapidement à toute situation d'urgence pour faire face à la précarité dans laquelle nos compatriotes peuvent tomber, lorsqu'aucun filet social n'est là pour les soutenir.

dépendante de sa capacité à exploiter et valoriser les atouts économiques, sociaux, culturels et humains dont il dispose. La présence de nos compatriotes français à l'étranger est l'une des conditions évidentes du rayonnement international de la France. La France rayonne à l'international grâce à cette présence française sur tous les continents. Nous avons une chance inouïe : c'est un magnifique réseau. Pour le général de Gaulle, la politique étrangère et donc, une certaine manière, la présence française à l'étranger était l'expression même de la Nation sur la scène internationale participer à la vie du milieu extérieur est pour toute nation plus qu'un droit, c'est un devoir, c'est l'expression normale de l'existence nationale. Il semble donc essentiel de soutenir et consolider ce réseau international de Français qui sont fondamentalement attachés à notre beau pays, la France. D'ailleurs, d'autres grandes puissances savent très bien soutenir

à nos compatriotes en Afrique, qui se trouvent dans des zones de conflit. Le contexte actuel de pandémie renforce également la nécessité de venir en aide à nos compatriotes à l'étranger. C'est la raison pour laquelle je voterai ce texte. L'amendement

portant sur la façon de répartir l'aide sociale : « J'ai été très surpris de constater que les élus consulaires n'ont pas été associés à la procédure d'aide sociale d'urgence accordée aux Français de l'étranger sans ressources. Ce dispositif annoncé le 30 avril marque la solidarité de la Nation avec nos compatriotes à l'étranger les plus fragiles. « À l'heure actuelle, les agents de l'administration consulaire attribuent cette aide sur leur seule évaluation. L'avis des élus est facultatif ou informel et leur rôle devrait se limiter à la possibilité de faire connaître ce dispositif. » En référence figure votre lettre, monsieur le secrétaire d'État, adressée aux parlementaires.

encadrer un peu plus la consultation préalable des conseils consulaires. Comme le disait l'un des brillants prédécesseurs de M. Le Drian,

il vaut mieux aider les gens qui ont des difficultés quand ils se tiennent encore debout et qu'ils savent que leurs revenus vont baisser, plutôt que d'attendre qu'ils ne soient à terre.

Finalement, les subventions accordées aux organismes locaux d'entraide et de solidarité sont évoquées en conseil consulaire et sont, à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE), sans que le conseil permanent pour l'action sociale puisse se prononcer. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la loi que les conseils consulaires seront consultés avant toute décision relative au versement d'une subvention de l'État versée à un organisme local d'entraide et de solidarité ou à un centre médico-social, particulièrement en période de crise. L'avis du conseil consulaire portera sur le montant et l'usage de la subvention de manière à éviter que ces subventions ne soient versées de manière discrétionnaire par la DFAE, sans avoir obtenu un avis précis et déterminé pour chaque subvention et pour chaque organisme local d'entraide et de solidarité. Quel est l'avis de la commission ? Tout d'abord,

tout à fait à la vocation de ces élus au suffrage universel direct que sont les conseillers consulaires. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

en lieu et place du gage habituel. En effet, plutôt que le gage classique consistant en une augmentation des droits et taxes sur les alcools et tabacs, nous avons recherché quelques idées, plus liées à l'international. Les différentes taxes sur l'aviation sont de vraies pistes, sans jeu de mots. sans jeu de mots. Nous avons donc été écologistes avant le résultat des élections municipales ; nous pensons qu'une augmentation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes serait opportune, d'autant plus qu'elle repose sur tous les gros avions, quelle que soit leur nationalité. L'intérêt d'une telle mesure réside dans le fait que l'État disposerait immédiatement d'un fonds pour intervenir, dans les plus brefs délais, en faveur des Français de l'étranger en temps de crise.

Nous nous sommes donc limités à la hausse de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Je ne voudrais